Monsieur le président,

les crédits des missions « Pouvoirs publics », « Conseil et contrôle de l'État » (et article 54 ), « Direction de l'action du Gouvernement » et du budget annexe « Publications officielles et information administrative

À cet égard, vous l'aurez remarqué, tant M. le président du Sénat que M. le président de l'Assemblée nationale ont marqué leur vive opposition

et que cette commission traiterait d'autres sujets connexes, annexes ou subséquents. On n'y comprend donc plus rien. Cela n'est ni clair ni acceptable.

de faire en sorte qu'il soit mis fin, purement et simplement, à cette mauvaise initiative qui consiste à créer une commission se substituant au Parlement, quels que soient, par ailleurs, la compétence, le talent et les convictions des personnes qui la composeraient. Acte vous est

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit qu'une mission spécifique regroupe les crédits alloués sous forme de dotations aux pouvoirs publics, dont le juge constitutionnel a rappelé le principe d'autonomie financière, qui relève de la séparation des pouvoirs. Ce budget est relativement constant depuis 2012, puisqu'il tourne autour de 1 milliard d'euros pour l'ensemble des institutions de la République.

Je regrette, à la suite de mon prédécesseur Jérôme Bascher, que ces financements extérieurs ne permettent pas d'appréhender la totalité des crédits dont dispose la présidence de la République et que devrait refléter la dotation.

De même, d'un point de vue interne, la réorganisation des services de l'Élysée, achevée en 2019, semble commencer à produire ses effets. Enfin, pour ce qui concerne l'exécution 2020, la crise sanitaire que nous traversons a conduit à une baisse des déplacements présidentiels, dont les crédits ont été réorientés pour financer des dépenses sanitaires et d'investissement. Malgré cela, l'exercice 2020 devrait être légèrement excédentaire. En ce qui concerne les dotations des assemblées parlementaires, elles sont stables, puisque gelées depuis 2012. concerne la Haute Assemblée, ce gel avait été estimé en 2020, à 388 millions d'euros, soit une somme supérieure à une année de dotation. Malgré une baisse des dépenses en 2021, la stabilité de la dotation conduit les assemblées à prévoir un nouvel important prélèvement sur trésorerie, qui permet de financer les dépenses d'entretien et d'investissement immobilier nécessaires au bon déroulement du travail parlementaire et à la préservation du patrimoine historique. Toutefois, comme mes prédécesseurs, j'appelle votre attention sur ce recours croissant aux réserves. Ces dernières vont s'amenuiser au fil des années, ce qui pose inévitablement la question de la soutenabilité de ce modèle à long terme. budget des chaînes parlementaires est stable. Il s'agit toutefois d'un sujet auquel je souhaite m'intéresser dans les prochains mois, en lien avec nos autorités et avec l'Assemblée nationale, car je sais l'importance de l'autonomie de chaque chambre en la matière.

Le budget du Conseil constitutionnel est relativement stable si l'on tient compte de la non-reconduction, cette année, du budget exceptionnel qui lui avait été affecté, en 2020, pour le contrôle de la première procédure de référendum d'initiative partagée relatif au fameux dossier d'Aéroports de Paris. Je salue la volonté du Conseil constitutionnel de mettre en place, dès 2021, en lien avec les juridictions, un véritable suivi de la question prioritaire de constitutionnalité, qui prend une importance significative, puisqu'elle représente désormais près de 80 % de son activité. Enfin, la dotation

au 12 novembre 2020, le nombre de plaintes était en augmentation, avec un total de 178 plaintes, dont 113 sont en rapport avec la covid. Pour 2021, cette hausse d'activité devrait se traduire par une augmentation des frais de justice, qui devrait néanmoins pouvoir être financée par un report des crédits de 2020. Il faudra toutefois demeurer vigilant quant aux frais éventuels générés par ce regain d'activité.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit un budget de

au programme « Conseil d'État et autres juridictions administratives ». Les juridictions administratives font face à une hausse considérable des recours.

la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a enregistré en 2019 le nombre de recours le plus important depuis sa création, avec 59 091 entrées enregistrées ; cela représente une augmentation de 40 % par rapport à 2018. Pis encore, la crise sanitaire a entraîné un nouvel allongement des délais de jugement, alors que ces derniers sont déjà supérieurs de près d'un mois aux délais inscrits dans la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.

Grâce à un important travail de réforme, le délai prévisible moyen de jugement devant les tribunaux administratifs a été divisé par deux en vingt ans, il convient de le souligner. cette dynamique vertueuse pourrait être interrompue par l'augmentation du contentieux. C'est pourquoi nous devons maintenir une vigilance particulière sur les délais de jugement des juridictions administratives au cours des prochaines années. Les crédits demandés pour la justice administrative augmentent de 2 %, sauf ceux qui sont accordés à la Cour nationale du droit d'asile. Cette évolution permettra de créer, en 2021, 29 emplois autorisés, destinés, d'une part, au renforcement des tribunaux administratifs, d'autre part, à la nouvelle cour administrative d'appel de Toulouse. Là encore, cette évolution me paraît non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. Je serai plus bref sur les crédits des autres programmes, qui, dans l'ensemble, évoluent peu par rapport à 2020. Le budget du Conseil économique social et environnemental (CESE) est stable en 2021, malgré le réel accroissement de son activité. Le CESE a bénéficié d'une augmentation de 10 % de ses crédits en 2020, afin d'organiser la Convention citoyenne pour le climat. En intégrant les moyens mobilisés par le CESE, le coût de l'organisation de cette convention s'est élevé

Le budget des juridictions financières demeure quasiment stable en 2021- on observe une légère augmentation de 0,3 % par rapport à 2020 -, malgré la création de 10 emplois supplémentaires, sur un total de 1 700 agents. Enfin, les crédits du programme 340, « Haut Conseil des finances publiques » augmentent de 213 % du fait du recrutement de cinq économistes supplémentaires.

Mes chers collègues, j'en ai terminé avec la présentation des crédits de cette mission, que je vous invite à adopter avec les modifications apportées par l'Assemblée nationale. Très bien

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission « Direction de l'action du Gouvernement » est l'une des rares missions budgétaires à ne pas être affectée par la crise sanitaire et économique que connaît notre

Cette hausse reflète les deux priorités stratégiques de la mission, qui font l'objet de moyens renforcés que nous saluons. La première priorité est le renforcement de la coordination interministérielle en matière de sécurité et de défense. L'actualité ne cesse d'en démontrer l'importance, en matière tant de lutte contre le terrorisme que de gestion de crise. L'action afférente, qui comprend notamment le budget du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), voit ainsi ses crédits augmentés de 9 millions d'euros. Cette hausse permettra notamment d'accompagner la montée en puissance de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), dont les effectifs seront renforcés de 40 agents à équivalent temps plein. La seconde priorité concerne la protection des droits et des libertés. Le budget qui nous est présenté prévoit ainsi le renforcement de plusieurs autorités administratives indépendantes exerçant leurs missions dans ce domaine, en particulier la Commission nationale de Ces dernières années, le législateur a étendu plusieurs fois le champ de compétences de ces autorités, qui ont connu une hausse considérable de leur activité. Le nombre de plaintes adressées à la CNIL a ainsi doublé en trois ans, tandis que le nombre de saisines du Défenseur des droits a augmenté de 50 % en cinq ans. Pour accompagner cette hausse, ces deux autorités indépendantes bénéficieront, en 2021, d'un renforcement bienvenu de leurs effectifs, à hauteur, respectivement, de 20 ETP et de 5 ETP. Si ces nouvelles

D'une part, certaines dépenses des services du Premier ministre, considérées comme exceptionnelles en 2020, n'ont pas été budgétées dans les crédits de la mission pour 2021, alors même qu'elles seront vraisemblablement reconduites. Il s'agit notamment des dépenses de communication du Gouvernement sur la crise sanitaire, qui s'élevaient à un total de 17 millions d'euros au 30 septembre 2020. Cette démarche consistant à occulter ces dépenses pour l'année 2021 a suscité des interrogations au sein de la commission des finances. D'autre part, certaines dépenses courantes des services du Premier ministre sont, quant à elles, présentées comme des dépenses exceptionnelles et figurent à ce titre dans le plan de relance, pour un montant total de plus de 500 millions d'euros. Il s'agit, par exemple, de dépenses destinées à renforcer la sécurité numérique de l'État ou à moderniser les postes de travail des agents publics. La majeure partie de ces dépenses ne présente, semble-t-il, qu'un lien ténu avec la relance économique du pays et aurait donc pu figurer dans les crédits de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ». Je terminerai mon propos par quelques mots sur le budget annexe « Publications officielles et information administrative qui connaît une forte baisse de ses recettes en raison du ralentissement de l'activité économique. Pour l'année 2021, les recettes du budget annexe s'élèveront ainsi à 159 millions d'euros, traduisant une baisse de 39 millions d'euros par rapport aux recettes perçues en 2019. Malgré ces prévisions en baisse, ce budget annexe pourrait dégager en 2021 un léger excédent, évalué à 6,7 millions d'euros et rendu possible par une nouvelle réduction des dépenses de personnel et de fonctionnement. Si cette érosion des recettes venait à se poursuivre, le modèle économique du budget annexe pourrait toutefois être durablement remis en cause. Telles sont, mes chers collègues, les différentes observations que je pouvais formuler au nom de la commission des finances. Au regard de ces éléments, celle-ci a décidé de proposer au Sénat d'adopter sans modification les crédits de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » et ceux du budget annexe « Publications officielles et information administrative ». La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec l'évolution technologique et la généralisation du numérique, la menace cyber ne cesse de se développer. La cybercriminalité s'est beaucoup professionnalisée et progresse à grande échelle grâce à des « rançongiciels » de plus en plus performants. Les organismes publics et les opérateurs critiques, comme les hôpitaux, ne sont désormais plus épargnés et l'on voit se multiplier les attaques contre les collectivités territoriales, qui commencent tout juste à prendre la mesure du problème. dit, les autres formes de cybermenaces, comme l'espionnage et les piratages, qui ciblent particulièrement les institutions et administrations publiques, progressent également. Il faut nous préparer aux cyberconflits de demain, qui sont déjà une réalité, sans bien sûr oublier les opérations de désinformation transitant sur les réseaux, qui cherchent à déstabiliser les démocraties, voire à déclencher des actes terroristes.

mais elle a aussi contribué à la prise en compte du risque numérique par les opérateurs privés et par les particuliers. Ainsi, l'Agence participe notamment au groupement d'intérêt public Action qui mène des actions tout à fait essentielles de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. À cet égard, je vous recommande la plateforme www.cybermalveillance.gouv.fr. ; vous y apprendrez les « gestes barrières » numériques, par exemple pourquoi et comment bien gérer ses mises à jour. En 2021, l'essaimage de l'Anssi au pôle cyber de Rennes et au campus cyber d'un immeuble de La Défense sera une contribution significative à la construction d'un écosystème français de la cybersécurité. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées se félicite des progrès considérables accomplis ces dernières années sous l'égide de l'Anssi. C'est en grande partie grâce à elle que, en matière de cybersécurité, la France fait partie des pays du premier cercle. Nous tenons toutefois à formuler deux recommandations. Malgré les avancées, les administrations publiques restent, dans l'ensemble, insuffisamment réceptives au risque cyber et ne prennent vraiment en compte celui-ci qu'après la survenue d'un problème majeur. Il est donc tout fait urgent d'appliquer la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, récemment refondue. En effet, celle-ci conforte le pilotage de l'Anssi sur les administrations et permettra, nous l'espérons, d'améliorer la diffusion des mesures préventives. Par ailleurs, nous recommandons d'accélérer la désignation des opérateurs de services essentiels afin d'étendre l'application de normes de cybersécurité à des activités ou fonctions qui, sans être critiques, sont pourtant essentielles à la vie de la Nation ; on perçoit bien, en ce La recrudescence actuelle des cyberattaques plaide en ce sens ; il s'agit bel et bien d'une course de vitesse. L'augmentation des crédits soumis à notre examen est le signe que cet enjeu important est bien pris en compte par le Gouvernement. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées s'est donc prononcée favorablement à leur adoption. Je rappelle

avis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon propos, complémentaire à celui de mon collègue Olivier Cadic, porte plus précisément sur la sécurité des réseaux mobiles de cinquième génération (5G). La commercialisation des offres 5G vient de démarrer la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a souhaité saisir l'occasion offerte par ce débat budgétaire pour faire le point sur l'application de la loi du 1 août 2019 sur la sécurité des réseaux mobiles. Cette loi confie à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dont nous examinons aujourd'hui les moyens budgétaires, le soin de délivrer aux opérateurs de télécoms les autorisations d'utiliser des équipements destinés à constituer leurs réseaux. Via les objets connectés, les réseaux de téléphonie mobile conditionnent le fonctionnement de notre économie et de notre vie quotidienne, ce qui est d'autant plus vrai en période de crise sanitaire. Ils doivent donc être tout à fait sûrs et protégés des interruptions de service. Un tel risque existe lorsque les équipements proviennent d'une entreprise étrangère soumise aux lois de son pays et aux éventuelles pressions de ses gouvernants. L'hypothèse d'un acte offensif étranger qui emprunterait ce canal est une menace majeure pour la sécurité de la Nation et doit être prise en compte.

Pour la commission des affaires étrangères et de la défense, le bilan est donc positif. Elle en prend acte et suivra attentivement les développements ultérieurs de ce dossier. Elle souhaite également insister sur la mise en place, à l'échelle européenne, d'une approche commune des risques de sécurité induits

de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je m'exprime donc au nom de Brigitte Micouleau, rapporteure pour avis. Chaque année, l'examen des crédits de la Mission interministérielle chargée de l'élaboration et du pilotage de la politique gouvernementale de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) nous donne l'occasion de faire un point sur les addictions dans notre pays. Dans un premier temps, la crise sanitaire n'a pas majoré les consommations de substances addictives, mais l'épidémie de covid-19, la crise économique et les angoisses qu'elles provoquent doivent nous inciter à redoubler de vigilance face aux risques de nouvelles addictions chez nos concitoyens les plus fragiles. Le tabac et l'alcool demeurent, en dépit de la diminution globale des usages, des tueurs en série responsables, respectivement, de 75 000 et 41 000 décès annuels. Il demeure nécessaire de faire reculer, par tous moyens, l'âge du premier usage. En matière de drogues illicites, la politique de réduction des risques et des dommages doit pouvoir s'appuyer, dans l'année à venir, et avant la fin de l'expérimentation, sur l'ouverture de nouvelles salles de consommation à moindre risque.

baisse est, toutefois, à mettre en perspective avec la mise en place du Fonds national de lutte contre les addictions qui favorise une coopération étroite entre les acteurs institutionnels engagés dans la lutte contre les conduites addictives. Doté de 115 millions d'euros et abondé, à partir de cette année, par les recettes liées à l'amende forfaitaire pour usage de substance illicite, le fonds garantit une plus grande efficacité de l'action publique. La Mildeca s'assure, par sa participation à ces instances de décision, de la cohérence entre les opérations de marketing social, programmées chaque année par Santé publique France, les dépenses de prévention de l'assurance maladie et les priorités gouvernementales de la politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Se fondant sur ce constat, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la Mildeca. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dois d'abord, s'agissant du budget de la Présidence de la République, informer le Sénat des conditions particulières dans lesquelles le rapporteur pour avis de la commission des lois a été conduit à rédiger son rapport. En effet, pour la deuxième année consécutive, M. le directeur de cabinet du Président de la République a refusé de me recevoir. Il a refusé de me recevoir, arguant de quelque prétexte qui, à mon sens, ne l'en empêchait nullement. Je répète

pays et la personne du chef de l'État, nous ne devons pas lésiner sur ces crédits de sécurité. Ceux-ci sont importants ; quand M. Strzoda me recevait, il me disait que le blindage d'une voiture coûte 800 000 euros.

avis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les juridictions administratives bénéficieraient, en 2021, d'une hausse de crédits de paiement de 2,7 % et d'un schéma d'emploi en augmentation de 28 équivalents temps plein C'est un renfort bienvenu, mais qui reste modeste au regard de la hausse importante du nombre d'affaires que les juridictions administratives enregistrent depuis plusieurs années. En 2019, l'augmentation des requêtes déposées devant les tribunaux administratifs est de 8,7 % et près de 6 % devant les cours administratives Parmi les contentieux traités par les juridictions administratives, le contentieux des étrangers a pris, au fil des ans, une place centrale. Il représente, en 2019, 51 % des affaires enregistrées dans les cours administratives d'appel et 41 % de celles enregistrées dans les tribunaux administratifs. Dans ces conditions, le défi reste le même : comment faire face, sans dégrader ni la qualité des décisions ni les délais de jugement ? Le Conseil d'État avance quelques pistes, notamment sur l'aide à la décision qu'il s'agirait de mieux mobiliser ou sur le développement de la médiation. Ces pistes ne semblent toutefois pas en mesure en 2021 ni même à moyen terme. Cette année encore, les performances des juridictions administratives reposeront avant toutes choses sur l'engagement individuel des personnels des juridictions administratives et sur leur sens du service public. Cette situation ne peut être pérenne et le programme 165 ne pourra pas échapper, selon moi, à un questionnement sur le renforcement des moyens humains et la revalorisation indemnitaire des personnels. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a atteint un pic historique, en 2019, en rendant 66 464 décisions. Les Les délais de jugement, qui avaient presque atteint l'objectif légal de cinq mois pour les formations collégiales en février 2020, à la veille du confinement, ont été fortement dégradés et sont désormais estimés à onze mois pour l'année 2020. Il est donc important d'accompagner la reprise d'activité de la CNDA dont la commission soutient la demande de report à l'année 2021 de la vingtaine d'emplois qui n'ont pu être pourvus en 2020 en raison de la crise sanitaire. Il s'agit d'une mesure Concernant Concernant le programme 164, « Cour des comptes et autres juridictions financières », les moyens prévus par le PLF pour 2021 seraient stables avec un schéma d'emploi prévoyant la création de 10 équivalents temps plein, dont 5 pour renforcer les fonctions de contrôle. Compte tenu de l'extension du périmètre des compétences des juridictions financières, la stabilité des moyens humains entraîne une nécessaire et toujours plus forte priorisation des contrôles des comptes et de la gestion. Or la baisse d'intensité des contrôles est une vraie question qui peut, à terme, entraîner une érosion de la confiance des citoyens envers leurs décideurs publics. Dans le cadre du chantier de réflexions stratégiques des juridictions financières « JF 2025 » lancé par le nouveau Premier président de la Cour des comptes, M. Moscovici, il me semble important de dégager, d'ores et déjà, quelques lignes de force. Il convient de conserver l'indépendance

pour une meilleure lisibilité des crédits alloués, il semble utile qu'une ventilation des crédits soit opérée entre la Cour des comptes et les CRTC, à l'instar de ce qui est fait dans le programme 165 entre le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.

mieux respecter la trajectoire de la loi de programmation militaire. Deuxième insincérité : le Gouvernement, nous semble-t-il, considère le plan de relance comme un supermarché où les administrations font leurs courses. Ainsi, 136 millions d'euros

d'un Haut Conseil pour le climat, dont on se demande à quoi il sert face au Conseil économique, social et environnemental ou au Haut-Commissariat au plan. La pandémie a conduit à une accélération de la révolution numérique, mais aussi à plus de vulnérabilité, compte tenu de la manière assez improvisée avec laquelle nous nous sommes tous mis aux visioconférences. C'est la raison pour laquelle il est absolument indispensable de soutenir l'évolution des crédits de l'Anssi.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette discussion budgétaire réunit trois missions qui, sans être les plus volumineuses de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021, revêtent une importance singulière. singulière. D'une grande diversité, ces crédits sont tous indispensables au bon fonctionnement de notre État de droit. Ils visent à garantir aux pouvoirs publics, aux organes chargés de leur contrôle ainsi qu'aux autorités indépendantes qui s'assurent du respect d'un certain nombre de libertés individuelles, les moyens nécessaires à leur action.

Une partie des crédits sera consacrée au financement de l'installation d'un site à Rennes, afin de constituer un pôle de compétence en matière de cyberdéfense. Cette nouvelle antenne permettra d'accueillir 200 agents. Je me félicite de l'ouverture de ces crédits indispensables pour notre stratégie en matière de cyberdéfense, enjeu ô combien essentiel en ces temps.

d'appel et de cassation. Cela mérite d'être souligné, car, en raison de la crise sanitaire, les indicateurs du délai moyen de jugement des affaires et la proportion de celles en attente se sont notablement détériorés. Il en sera, sans aucun doute, de même au début de Je souhaite donc saluer le renforcement des effectifs dans les juridictions administratives, puisque 28 ETP supplémentaires viendront grossir leurs rangs. Quant aux juridictions financières, Quant aux juridictions financières, elles gagneront 5 ETP, ce qui permettra, notamment, de préparer le mandat de de la Cour des comptes en tant que certificateur des comptes de l'ONU pour la période 2022-2028. En effet, la Cour des comptes et les juridictions financières ont moins souffert des conséquences de la crise sanitaire, puisque leurs modes de fonctionnement sont davantage dématérialisés. Leurs crédits sont en légère progression, notamment sous l'effet de schémas d'emploi positifs. Cette augmentation conduira à 10 recrutements supplémentaires en 2021, hausse qui s'inscrit dans la tendance de l'année passée. Concernant le CESE, son budget se stabilise à l'approche d'une réforme majeure. La réduction du nombre de membres du CESE permettra une baisse des dépenses liées aux indemnités des conseillers économiques permettant de absolument nécessaires pour mettre en oeuvre ses nouvelles prérogatives, notamment en matière de participation citoyenne. Pour ces raisons, le groupe Les Indépendants votera les crédits de ces trois missions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'ensemble des crédits que nous examinons cet après-midi me permet d'intervenir sur plusieurs questions qui concernent le coeur de l'État, le système de commandement

Chaque ministère n'a pas la force de travail ni les équipes permanentes aptes à produire une étude d'impact globale, et forcément pluraliste, sur chaque sujet abordé.

devrions travailler. Les autorités administratives indépendantes, du point de vue de leur gestion, méritent un témoignage de satisfaction. Les regroupements qui pouvaient être faits l'ont été.

sauf la CNIL, constituent des employeurs de petite taille. Il me semble que la synergie entre la direction de la fonction publique, au niveau central, et les autorités administratives indépendantes pourrait être améliorée dans le sens d'une continuité de carrière. On

du nombre des dossiers dont sont saisies les juridictions est en grande partie liée au contentieux des étrangers, lequel a fait l'objet d'adjonctions et de modifications de procédure, souvent un peu improvisées au cours des dernières années. Un rapport du Conseil d'État préconise un certain nombre de

trois remarques. Premièrement, le tout sécuritaire est affiché tel quel dans les priorités où la sécurité figure en pole position. C'est sans doute justifiable pour ce qui est du renforcement des moyens du GIC ou de l'Anssi et de la création à venir d'une antenne à Mais c'est sous cette injonction du tout sécuritaire que la Miviludes a été transférée au ministère de l'intérieur. Nous continuons à penser que cette décision est regrettable. Il va de soi que cette mission interministérielle relève, par essence, de bien d'autres problématiques que celles de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Nous pensons notamment aux domaines de l'éducation ou de la santé. de décès liés à l'alcool ou au tabac, ainsi que celui des consommateurs de substances psychoactives et de nouveaux produits tels que la kétamine ou le protoxyde d'azote, continue d'être très important. En outre, les confinements et la crise que nous vivons ont tendance à augmenter ces conduites addictives.

Deuxièmement, s'agissant de la mission « Conseil et contrôle de l'État », nous déplorons le traitement réservé par le Gouvernement à la Cour nationale du droit d'asile. Depuis trois ans, nous rappelons qu'il ne peut y avoir de République sans politique humaniste du droit d'asile, qui passe par un accueil digne et sécurisé des réfugiés dans notre pays. Or, dans la série des ordonnances prises dans le cadre de la crise sanitaire, celle du 13 mai dernier prévoit que, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, la Cour peut statuer sur tous les dossiers en audience à juge unique et avec un recours accru à la vidéo-audience. Cela nous inquiète fortement. Même si le Gouvernement a été désavoué par le Conseil d'État, nous savons qu'il entend poursuivre sa politique comptable en la matière. Cette volonté ne sera pas sans conséquence sur le nombre de reports de procédures et sur l'explosion à venir

Après la crise des « gilets jaunes », le Président de la République a demandé à des citoyens tirés au sort, de travailler pour formuler des propositions ambitieuses sur le climat, avant de les recevoir à l'Élysée pour annoncer qu'il s'engageait à faire passer en conseil de défense écologique ou à soumettre au Parlement toutes leurs propositions. l'a pas empêché d'en élaguer quelques-unes, notamment la taxe de 4 % sur les dividendes ... Les mois qui ont suivi ont prouvé l'inverse, laissant place à l'immobilisme, voire à certains reculs sur les propositions. Après avoir étouffé la soif d'égalité républicaine des quartiers populaires par l'enterrement en première classe du plan Borloo, le cri de la justice sociale et fiscale des « gilets jaunes » avec le grand débat national, qui n'aura débouché sur rien, ... Oui ! ... vous vous apprêtez, monsieur le en dénaturant les propositions de justice climatique de la Convention citoyenne. C'est vrai qu'il est compliqué pour un gouvernement de reconnaître le crime d'écocide alors que, en même temps, il réintroduit les néonicotinoïdes ! Ce déni de démocratie

Toutes ces questions, mais surtout les orientations choisies par le Gouvernement dans la gestion de ses politiques publiques, nous conduisent à voter contre les budgets de ces trois missions. La parole est

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais m'attacher à faire quelques remarques sur les missions « Direction de l'action du Gouvernement » et « Conseil et contrôle de l'État Tout d'abord, la mission « Direction de l'action du Gouvernement » connaît une nouvelle fois une modification de son périmètre d'action, avec la création d'un nouveau programme dont l'objet est de financer la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, avec un engagement financier important dès 2021. Dans la continuité des budgets précédents, on note un renforcement des moyens dévolus à la lutte contre le terrorisme, aux moyens des services de renseignement et à la coordination des services de sécurité et de défense nationale. Ainsi, nous tenons à saluer la hausse des moyens alloués à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il convient par ailleurs de saluer les efforts consentis en matière de recrutement dans les différentes organisations publiques, notamment la CNIL, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi que le Défenseur des droits. Ces instances jouant un rôle majeur de protection des libertés dans notre système démocratique, l'augmentation de leurs moyens est la bienvenue. Cela étant, nous pouvons nous interroger sur la sincérité budgétaire des crédits attribués au service d'information du Gouvernement.

force est de constater que l'on s'y perd un peu entre les actions qui passent d'un ministère à l'autre. À ce propos, je souhaite répéter les regrets que nous inspire le transfert de la Miviludes au ministère de l'intérieur. Cet organisme, dont les moyens ont été réduits, risque de perdre sa spécificité au profit des moyens dévolus à la lutte contre la radicalisation. concerne la mission « Conseil et contrôle de l'État », il me paraît important de souligner la nécessité de recourir à des moyens humains adaptés afin d'assurer la qualité du travail des juridictions administratives. Si l'on peut se satisfaire de la hausse des crédits de paiement, malgré une baisse importante des autorisations d'engagement, ces crédits permettront essentiellement de mettre en oeuvre les projets immobiliers des juridictions administratives et, dans une moindre mesure, de renforcer leurs effectifs pour faire pour faire face à l'augmentation du contentieux dans les tribunaux administratifs. Même s'ils tendent à diminuer depuis 2002, les délais de jugement restent la préoccupation majeure des juridictions administratives. En 2021, du fait de l'état d'urgence sanitaire, les délais de jugement vont se dégrader. Cette situation a des conséquences particulièrement dramatiques, notamment pour les justiciables de la Cour nationale du droit d'asile. celle-ci n'a pas pu effectuer les recrutements nécessaires à son activité. À cet égard, une augmentation plus importante des autorisations d'engagement et des crédits de paiement aurait été appréciable. Au vu du contexte international que nous connaissons, qui a un impact sur le nombre de demandeurs d'asile, la réduction des délais de recours et l'accélération des procédures devant la CNDA entraînent une surcharge de travail et ne permettent pas un accompagnement correct des personnes. Nous devons être particulièrement vigilants, afin que l'État de droit ne puisse être remis en cause. L'année 2021 devrait être marquée par la mise en place de la réforme du Conseil économique, social et environnemental, adoptée au mois d'octobre 2020 et dont les décrets d'application devront être publiés avant le 1 juin 2021. Rappelons que le CESE est la troisième assemblée de la République. Il est à l'origine de nombreux projets. Il a notamment été chargé d'organiser la Convention citoyenne pour le climat. La réforme envisagée vise à faire du CESE une instance consultative de premier ordre. Elle prévoit notamment la possibilité d'organiser des consultations publiques et de rendre des avis sur la mise en oeuvre de lois traitant de sujets économiques, sociaux et environnementaux, sur demande du Gouvernement ou du Parlement, la faculté d'associer à ses travaux des conseils consultatifs de collectivités locales, des composantes de la société civile et des personnes tirées au sort. Bien que cette réforme prévoie la réduction du nombre de membres du CESE, il est surprenant que le budget alloué soit stable par rapport à 2020. Eh oui ! En effet, le renforcement de ses missions implique un accroissement significatif de la charge de travail et nécessiterait donc des moyens plus importants.

: bien des actions qui relèvent de ces budgets se retrouvent, en fait, dans le plan de relance. Cela nuit grandement à la lisibilité des programmes, et donc à l'action publique.

En revanche, concernant la mission « Conseil et contrôle de l'État », nous considérons que la prise en compte des missions de la CNDA est insuffisante. Nous nous abstiendrons donc sur les crédits de cette dernière mission. La parole

feu le référendum d'initiative populaire sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Il me semble que cette privatisation n'est plus totalement à l'ordre du jour

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les juridictions administratives et financières et ne m'attarderai pas non plus sur les programmes de la mission « Pouvoirs publics Je mettrai plutôt en exergue quelques points qui me paraissent révélateurs des priorités données par le Gouvernement dans sa conduite de l'État. Les crédits alloués à la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives se révèlent très insuffisants : l'action correspondante est la seule à ne pas bénéficier d'une augmentation de ses crédits sur l'année 2021. Les budgets alloués au Défenseur des droits ainsi qu'au Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont eux aussi insuffisants : ces deux institutions fondamentales pour le contrôle et la protection des libertés individuelles devraient bénéficier de conditions matérielles améliorées. Le Défenseur des droits a connu une augmentation de 40 % de ses saisines entre 2014 et 2020 et devrait être soutenu dans la nécessaire déconcentration de son activité et dans le renforcement de son réseau de délégués territoriaux. Notre groupe présentera deux amendements tendant à augmenter les moyens humains et matériels de ces deux institutions. Et que dire de la façon de traiter l'urgence climatique ? Le jeune Haut Conseil pour le climat devrait être une instance utile dans ce cadre. Il a dénoncé, pas plus tard que mardi, le retard considérable de la France dans la rénovation énergétique des bâtiments.

je partage ce qu'ont dit certains de mes collègues. Je prends acte que les crédits « permettront d'organiser une nouvelle Convention citoyenne ou d'associer la parole citoyenne », notamment par la mise en place de pétitions dématérialisées. Nous sommes favorables à l'allocation de crédits pour stimuler ces nouvelles formes d'expression, que nous estimons revitalisantes pour notre démocratie. Toutefois, un doute m'envahit, non sur la pertinence de tels travaux, mais sur le manque de prise en compte et de mise en oeuvre de leurs conclusions par votre gouvernement.

qu'on le veuille ou non, un afflux plus important de demandeurs dans les prochaines années. Accueil des migrants, contrôle et protection des libertés individuelles, urgence climatique, prise en compte de la participation citoyenne

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le contexte sanitaire et sécuritaire actuel nous appelle à porter une attention particulière aux crédits des missions budgétaires que nous nous apprêtons à examiner. En effet, ayant pour vocation de financer une grande partie de notre structure institutionnelle, ces missions combinent à la fois des objectifs de bon fonctionnement de la justice, de contrôle de notre administration et de confiance en l'action publique. Alors que l'obscurantisme nous met au défi, nous avons le devoir de défendre avec vigueur notre modèle de société, à la fois démocratique, ouverte, mais aussi inflexible avec l'intolérance. Par ailleurs, face à une crise sanitaire dont nous sommes loin d'être sortis, il faut toujours rappeler que la première cause de l'État est de protéger ses citoyens, notamment en garantissant le respect de l'ordre public dans sa dimension sanitaire. Loin des fantasmes délirants des complotistes ou de l'absence de sens civique des plus irresponsables, nous devons, en tant que législateurs, donner aux pouvoirs publics comme aux organes chargés de leur contrôle tous les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. La crise sanitaire a notamment conduit de nombreux fonctionnaires à travailler différemment, souvent à distance, en s'adaptant à ces nouvelles contraintes. Je tiens évidemment à saluer leur engagement et leurs efforts dans ce contexte difficile.

va bénéficier d'une réforme importante, dont l'objectif est de mieux prendre en compte la parole citoyenne dans le débat public. Partisan, à titre personnel, de la démocratie participative, je ne peux qu'encourager cette réforme,

Avec cet exemple, mes chers collègues, je veux vous faire prendre conscience que l'insularité doit évidemment être prise en compte. J'espère que le Sénat reviendra sur ce sujet. La crise sanitaire a eu et continue d'avoir des conséquences importantes sur l'activité des juridictions administratives et financières. Les stocks et les délais de jugement se sont évidemment dégradés, alors que la juridiction administrative avait entrepris et réussi, depuis plusieurs années, une politique ambitieuse de modernisation de son organisation et de ses méthodes de travail. Malgré tout, je me félicite de la formidable capacité d'adaptation à une situation inédite dont la juridiction administrative a su faire preuve et note une évolution positive des crédits de paiement, Concernant la mission « Direction de l'action du Gouvernement », il faut se réjouir du renforcement des moyens alloués à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dont une partie des crédits seront consacrés au financement de l'installation d'un site à Rennes, afin de constituer un pôle de compétences en matière de cyberdéfense. C'est une bonne nouvelle pour notre stratégie en matière de cyberdéfense, outil indispensable de la lutte que mène notre pays contre le terrorisme. Cela reflète également la prise de conscience que la criminalité s'est emparée de l'outil numérique pour rançonner ses victimes. Nos concitoyens exigent à bon droit que leurs élus soient irréprochables, alors que toute crise sociale entraîne son lot d'antiparlementarisme et de populisme. Prenons donc garde non seulement à maintenir les exigences de probité, mais encore à faire savoir que nous le faisons. La crise du covid-19 a aussi eu un impact sur l'organisation des travaux parlementaires : nous avons dû nous adapter à de nouvelles méthodes de travail.

de la lutte contre les dérives sectaires. Je crains par conséquent que nous n'ayons à constater, malgré la volonté du Gouvernement, un affaiblissement de l'action de l'État sur ce sujet. Le groupe du RDSE votera néanmoins les crédits de cette mission.

apprécie l'effort budgétaire qui est réalisé en direction de la CNIL pour la doter de moyens supplémentaires, car on voit bien que le renforcement de la réglementation, notamment

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

ainsi que par les rapporteurs pour avis, qui ont, comme chaque année, produit une analyse exigeante et précise des crédits sur lesquels le Sénat doit se prononcer aujourd'hui. À titre liminaire, je rappellerai, comme certains l'ont déjà souligné, que la crise sanitaire a obligé l'ensemble des personnels relevant des missions que nous examinons à travailler différemment, souvent sous des contraintes difficiles, à distance, en s'adaptant dans l'urgence à des méthodes nouvelles. Je voudrais ici saluer leur engagement et les efforts qu'ils ont fournis pour assurer la continuité des missions importantes qui leur sont confiées. Permettez-moi à présent d'entrer un peu plus dans le détail des crédits qui vous sont présentés et de répondre, dans la mesure du possible, à certaines de vos interrogations.

République font l'objet d'une analyse détaillée sur la base des questionnaires parlementaires de l'ensemble des rapporteurs et des entretiens avec les rapporteurs spéciaux, conformément à l'article 57 de la loi organique

et le prélèvement sur disponibilités, qui fait souvent l'objet de vos attentions, est en baisse pour atteindre 2,5 millions d'euros. Ces moyens illustrent les effets positifs de la réorganisation des services de la présidence,

l'Élysée entreprend des travaux de renforcement de sa sécurité, notamment de ses systèmes d'information, ce qui apparaît pour le moins nécessaire dans le contexte de menace terroriste et de tensions géopolitiques

de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui permettra de mieux connaître son usage, dix ans après son instauration. Monsieur Laménie, je me permettrai de m'abstenir de tout commentaire concernant le budget de votre assemblée. Il n'appartient pas au Gouvernement, au nom de la séparation des pouvoirs, d'apprécier le niveau de la dotation des assemblées parlementaires. La crise sanitaire a donné lieu à un certain nombre de plaintes devant la Cour de justice de la République, ce qui a pu conduire à s'interroger sur le niveau de sa dotation. Comme l'ont indiqué vos rapporteurs, cette hausse de l'activité sera financée par le report du solde de la dotation non consommée en 2020, avec l'accord du ministère de l'économie, des finances et de la relance. La mission « Conseil et contrôle de l'État » retient, comme chaque année, l'attention de l'ensemble des Ces crédits, en hausse de 2 %, traduisent un effort constant d'accroissement de la masse salariale et d'investissement depuis le début du quinquennat. Le PLF pour 2021 s'inscrit dans la trajectoire d'accroissement des moyens humains des juridictions administratives avec la création de 28 postes, notamment au bénéfice de la nouvelle cour administrative d'appel de Toulouse qui verra le jour en 2022. Cette augmentation des moyens, saluée par MM. Richard et Menonville, s'avère indispensable pour faire face à la hausse importante des contentieux, comme l'a souligné votre rapporteur spécial, M. Bilhac. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui a bénéficié de 80 % des créations d'emplois dans les juridictions administratives depuis cinq ans, soit 375 ETP, a particulièrement souffert de la période de confinement et de la crise sanitaire en général, comme l'ont rappelé MM. Benarroche et Gay. Je salue, dans la lignée des propos tenus avant moi, le report sur l'année 2021 des créations de postes qui n'ont pu intervenir en 2020 pour les raisons que vous connaissez, afin de poursuivre nos efforts visant à garantir l'effectivité du droit d'asile. Si la situation sanitaire le permet, la CNDA devrait pouvoir se rapprocher de sa capacité de jugement maximale au cours de l'année 2021 et tendre vers les objectifs prévus par la loi. Le fonctionnement de la Cour des comptes et des juridictions financières appelle moins de commentaires. Elles bénéficient cette année d'un schéma d'emploi positif qui conduira à dix recrutements supplémentaires en 2021. La hausse des crédits de personnel du Haut Conseil des finances publiques suscite des interrogations dont nous reparlerons. L'Assemblée nationale a ainsi adopté un amendement afin de limiter cette hausse à deux emplois. Le Haut Conseil pourra toutefois effectuer des recrutements supplémentaires afin d'exercer au mieux sa mission d'expertise indépendante tant auprès du Gouvernement que du Parlement. En dépit de ces recrutements, le Haut Conseil demeurera sur la scène européenne une institution budgétaire indépendante de taille très réduite. Enfin, le Conseil économique, social et environnemental conserve un budget stable. La réforme, en cours d'examen devant le Parlement, permettra de rénover le fonctionnement du CESE tout en garantissant la juste représentation des territoires- nous sommes sensibles à cette question. La réduction du nombre des membres du CESE permettra de dégager les économies nécessaires pour mettre en oeuvre les nouvelles prérogatives du Conseil, notamment en matière de participation citoyenne.

de l'action du Gouvernement » à laquelle est adjoint, pour 2021 et 2022, un nouveau programme consacré à la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Si l'on isole les crédits de ce programme éphémère, les crédits de la mission progressent de 2,7 en 2021. La hausse des crédits du programme « Coordination du travail gouvernemental » vient renforcer la coordination interministérielle en matière de sécurité et de défense. Le secrétariat général de la défense comme l'ont souligné votre rapporteur spécial Paul Toussaint Parigi ainsi que l'ensemble des rapporteurs. L'Anssi fait l'objet d'une attention particulière de MM. Cadic, Vallet et Richard qui soulignent sa grande compétence, comme en atteste sa forte attractivité. La création d'un pôle cyber à Rennes devrait y contribuer

Durant la crise sanitaire, ce service a notamment été chargé d'une plateforme téléphonique d'information des citoyens qui a engendré un coût important, de l'ordre de 8,5 millions d'euros, auquel se sont ajoutées des dépenses supplémentaires de communication. Nous pouvons espérer que le

Comme l'an dernier, un certain nombre de créations d'emplois et de missions concernent le programme « Protection des droits et libertés » et visent à permettre aux autorités administratives indépendantes d'exercer au mieux leurs prérogatives. Je rejoins ceux qui, comme MM. Leconte et Canevet, saluent le schéma d'emploi dynamique qui bénéficiera en particulier à la CNIL, avec la création de vingt postes pour accompagner la mise en oeuvre du RGPD, même si j'ai bien noté les points de vigilance à retenir. Le nouveau programme de la mission, qui permettra l'organisation de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, représente un budget total de 150 millions d'euros sur deux ans, ce qui correspond à peu près aux dépenses constatées lors du dernier exercice, en 2008, dont 47,4 millions d'euros de crédits de paiement en 2021 pour les réservations et opérations de communication en amont de la présidence.

raison, monsieur le ministre.

et techniques, mais à la mise en place, par les administrations compétentes, d'un suivi exhaustif de ce phénomène. Au demeurant, la Cour, qui se situe à équidistance du Parlement et du Gouvernement, arrête librement et en toute indépendance sa programmation, comme le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de le rappeler.

Conseil pour le climat fait l'objet d'un nombre croissant de saisines, ses moyens sont restés constants depuis sa création en 2019 par le Président de la République. Le Haut Conseil dispose, à l'heure actuelle, d'un budget de fonctionnement de 500 000 euros et de 6 équivalents temps plein, contre 24 pour son homologue britannique, comme cela a été dit.

dans le débat public, la question du renforcement des moyens financiers et humains du Haut Conseil pour le climat doit donc être posée. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement ; quant à moi, à titre personnel, j'y suis favorable.

à disposition du Haut Conseil ses moyens administratifs et financiers- il faut quand même le souligner -, lesquels sont mutualisés avec l'ensemble des organismes qu'il coordonne. Cela paraît suffisant ! Le HCC peut en outre mobiliser l'ensemble des experts et des organismes publics intervenant dans le domaine du climat,

le HCC- vous l'avez dit -est désormais une autorité installée dont les travaux sont reconnus. Il remplit donc la mission voulue par le Président de la République, qui était de créer un organisme chargé d'apporter un éclairage indépendant et neutre sur la politique du Gouvernement pour la lutte contre le changement climatique et sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux vous gagez votre amendement par la réduction des crédits de la présidence française de l'Union européenne, alors même que celle-ci sera l'occasion de porter au niveau européen l'ambition de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Avis défavorable.

peut-être le Royaume-Uni ne dispose-t-il pas d'un office parlementaire chargé de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques analogue à celui qui existe en France, avec 18 députés, 18 sénateurs,

Nous avons un Conseil économique, social et environnemental dont nous déplorons qu'il ne soit pas utilisé comme il faut. Or il a aussi cette compétence environnementale. Eh oui ! Je rappelle que le Haut Conseil pour le climat

Pour des raisons de cohérence et de simplification, il est donc préférable de s'appuyer sur le CESE plutôt que de renforcer cette petite structure

Il doit donc assurer un meilleur maillage territorial en renforçant son réseau de délégués territoriaux- tel est l'objet de cette augmentation de moyens. En outre, depuis peu, le Défenseur des droits s'est attelé à un nouveau sujet : je je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore noté, qu'il est chargé de la protection et de l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Il a ainsi été saisi de 84 dossiers en la matière en 2019. Pour poursuivre ses travaux dans ce domaine, le Défenseur des droits se doit de recruter une équipe spécialisée. Les besoins ont été évalués à 10 ETP supplémentaires

Comme cela a été dit, la version initiale de cet amendement avait pour objet une hausse de 2 millions d'euros, soit 9 % du budget total du Défenseur des droits. Ce montant apparaissait disproportionné à la commission des finances au regard du souci de maîtrise globale de la dépense publique.

Le PLF pour 2021 prévoit d'ailleurs une augmentation des moyens alloués à ce réseau en permettant d'accroître de 20 le nombre de délégués territoriaux, passé- je le rappelle -de 398 en 2014 à 520 en 2020 grâce à une hausse des crédits affectés à leur indemnité représentative de frais. En conséquence, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dotation et les moyens budgétaires attribués au Défenseur des droits, qui sont de 23 millions d'euros et ont été alloués pour lui permettre l'accomplissement de ses missions.

Il y a deux ans, le Gouvernement a élaboré un plan national de lutte contre les addictions sur cinq ans. Ce plan compte 6 axes, 19 priorités et 200 mesures mises en oeuvre par différents ministères et par différents opérateurs, associations et organismes. Dans ce plan, il faut distinguer l'esprit et la lettre. Le Gouvernement confie à la Mildeca des objectifs d'envergure, afin de répondre à des enjeux sociaux, sociétaux et surtout de santé publique considérables- cela a été dit en discussion générale -, tout en diminuant les moyens qui

On nous dit que les moyens sont redéployés : ici un fonds de lutte contre les addictions aux substances psychoactives porté par l'assurance maladie, là des moyens transférés au ministère de l'intérieur pour l'Office

Pourtant, s'agissant de la lutte contre les addictions, la tâche demeure immense. Les campagnes de sensibilisation et d'information ont porté leurs fruits sur la consommation d'alcool et de tabac, mais les bouleversements profonds du quotidien, provoqués notamment par le premier confinement, démontrent que les avancées sont fragiles. De récentes études ont montré que la consommation de tabac, d'alcool et de drogues, ainsi que le recours à des substances psychoactives

La baisse de 357 000 euros par rapport à 2020, à laquelle font référence les auteurs de l'amendement, correspond en réalité à une simple mesure de transfert, les missions du Centre interministériel de formation anti-drogues ayant été transférées au ministère de l'intérieur. À périmètre constant, c'est-à-dire corrigé de cette mesure de transfert, les moyens de la Mildeca sont parfaitement stables par rapport à la loi de finances pour 2020. Cet amendement me semble donc sans objet ; la commission demande à ses

et confisqués. De surcroît, en plus des crédits sur lesquels vous êtes appelés à délibérer cet après-midi, elle aura bénéficié, en 2020, de crédits supplémentaires à hauteur de 2,5 millions d'euros. Une stabilité des dotations à

à cet égard, nous connaissons le travail des services de la police, de la gendarmerie et des douanes -, mais aussi prendre en charge les personnes qui sont complètement cassées, abîmées, par ces fléaux.

Le CGLPL est une autorité administrative indépendante qui a pour mission de veiller à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité. Cette institution est fondamentale, parce qu'elle opère un contrôle de tous les lieux de privation de liberté, des centres de rétention administrative aux hôpitaux psychiatriques en passant par les locaux de garde à vue et les établissements pénitentiaires. Ses recommandations sont essentielles dans ces lieux où les citoyens n'ont aucun droit de regard. Compte tenu par ailleurs des récentes condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, sanctionnant la densité carcérale des maisons d'arrêt

l'amendement n° II-685 rectifié. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits. Nous allons aux voix ces crédits. Nous allons procéder au vote des crédits du budget annexe « Publications officielles et information administrative », figurant à l'état C. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits. Nous avons achevé

de la hausse quasi ininterrompue de ces crédits depuis 2010. Cela concerne donc au moins deux gouvernements. D'où provient cette augmentation ? C'est simple, elle provient d'abord des remboursements de crédits de TVA, la part la plus importante des remboursements et dégrèvements d'impôts avec 56,6 milliards d'euros. En sept ans, la sous-action relative aux restitutions de TVA a augmenté de 14,2 milliards d'euros. Dès lors, madame la ministre, il est inutile de vous préciser que je considère comme absolument nécessaire

et comment cette priorité est-elle gérée par le Gouvernement, madame la ministre ? Une action résolue permettrait de dégager de nouvelles ressources publiques, ce qui nous éviterait, par exemple, d'être suspendus à la décision de l'Union européenne de subventionner le plan de relance ! Lors des débats sur ce PLF pour 2021, j'ai aussi largement défendu la baisse des taux de TVA concernant les produits et les services essentiels aux personnes et à leur dignité.

Le coût de ce dispositif reste éminemment considérable pour les finances publiques, après avoir atteint quasiment 20 milliards d'euros en 2019. Inutile de mentionner le rapport éloquent de France Stratégie sur le sujet, largement cité dans l'hémicycle.

ils permettent à l'administration d'accorder au contribuable une minoration du montant des pénalités dues, mais également des droits demandés. Cette pratique est utilisée lors de redressements complexes, notamment en matière de fiscalité internationale. Sur les 116 règlements d'ensemble opérés en 2019, portant sur une remise totale 1,6 milliard d'euros, les droits ont été minorés de 1,12 milliard d'euros.

Dans cette affaire, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Paris avaient donné raison à l'entreprise au motif que « la société Google Ireland Limited ne dispose pas en France d'un établissement stable, au sens de la convention franco-irlandaise

programme s'effondrent, puisqu'ils passent de 23 milliards d'euros à 7 milliards d'euros. Deux événements expliquent cette contraction. D'abord, la réforme de la taxe d'habitation et, ensuite, la réforme des impôts de production. la réforme de la taxe d'habitation, il est utile de se rappeler que nous arrivons, en 2021, dans la deuxième phase de la réforme. Jusqu'ici, l'allégement introduit en loi de finances pour 2018 avait pris la forme d'un dégrèvement et, par voie de conséquence, son coût était retracé par la mission dont je rapporte les crédits. ce dégrèvement s'était ainsi traduite par une hausse importante des crédits de la mission : 3 milliards d'euros supplémentaires en 2018, 6 milliards d'euros supplémentaires en 2019 et 14 milliards d'euros supplémentaires en 2020. À compter de 2021, ce dégrèvement est transformé en exonération et le produit de la taxe d'habitation est perçu par l'État.

La politique, c'est l'art de chercher les problèmes, de les trouver, de les sous-évaluer et ensuite d'appliquer de manière inadéquate les mauvais remèdes. » Il s'agit, bien

bien pire ! J'en veux pour preuve la gestion des billets de trésorerie. Au moment où la France allait un petit peu mieux, elle a su diminuer son stock de billets de trésorerie pour, le moment venu, pouvoir émettre beaucoup de dette

a eu lieu en 2011. En 2011, la France n'a pas infléchi sa trajectoire de dette. Depuis, elle n'a fait qu'augmenter toute seule, négligemment. Ce n'était pas important parce que les taux baissaient. Nous avons connu ce paradoxe incroyable qui a consisté à multiplier par deux notre dette par rapport au PIB

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, le temps m'étant compté, je retiendrai trois points principaux de mon exposé. un élément de contexte. En 2020, la donne a sensiblement changé pour l'État actionnaire et sa doctrine. Telle la marée, l'ambition de 2017 a reflué. En prenant les commandes, le Gouvernement a redéfini les contours de sa doctrine : les participations de l'État étaient conçues comme un placement « à la papa lequel ne saurait échapper à la disruption en vogue à l'époque. Pour cela, un mouvement de « respiration » du portefeuille a été engagé, ce qui s'est concrétisé par la cession de la Française des jeux. La privatisation d'Aéroports de Paris devait suivre. Trois ans plus tard, « nouveau monde » accuse ses premières rides : à l'aune des événements exceptionnels que nous traversons, le Gouvernement a infléchi sa doctrine. Derrière cet élément de langage, c'est en réalité au retour de la conception qui prévalait jusqu'alors que nous assistons, avec la mobilisation de la prise de participation publique comme levier de politique économique. Je ne peux qu'approuver ce retour à la raison je suis convaincu que l'intervention en capital de l'État- je dis bien en capital -permet d'apporter une réponse, en soutien de nos entreprises, de nos savoir-faire et de nos emplois. Toutefois, je m'étonne de constater la très faible consommation des 20 milliards d'euros de crédits exceptionnels ouverts dans le deuxième collectif budgétaire, puisque seulement 20 % d'entre eux ont été consommés. Malheureusement, la sincérité budgétaire semble faire partie des « victimes collatérales » de la crise sanitaire. M. Martin Vial, commissaire aux participations de l'État, m'a indiqué qu'une recapitalisation de la SNCF devait intervenir avant la fin de l'année,

comment expliquer cette situation ? Vous parlez d'une doctrine « infléchie », mais c'est plutôt le constat d'un État actionnaire « à genou » qui s'impose. Deuxième point de mon exposé, ce constat ne peut qu'être renforcé par le dossier de la rentrée, qui continue de faire grand bruit et nous inquiète sur toutes les travées. Je parle, bien évidemment, de l'acquisition de Suez par Veolia. S'il s'agit d'une affaire entre entreprises à capitaux privés, l'État actionnaire est indirectement concerné au titre de la participation qu'il détient dans Engie. Or, lors du conseil d'administration du 5 octobre dernier, l'État a été mis en minorité sur le vote de la résolution concernant l'offre d'acquisition par Veolia des 29,9 % du capital de Suez détenus par Engie. au-delà des appréciations personnelles que nous pouvons avoir sur l'opportunité de la fusion, c'est bien la façon dont l'État actionnaire a appréhendé le dossier qui suscite mes interrogations. En effet, l'État a, sinon suggéré, du moins avalisé dès le premier semestre la décision d'Engie de recentrer ses activités et, partant, de mettre en vente sa participation au capital de Suez. C'est pourquoi, madame la ministre, la surprise invoquée ne saurait justifier l'attentisme de l'État actionnaire face à l'offre de Veolia. Mes chers collègues, sachez que le Gouvernement s'est montré, jusqu'à présent, peu coopératif. Non seulement Bruno Le Maire a perdu le chemin du Sénat, mais figurez-vous que son cabinet a décliné ma demande d'audition, jugeant que tel n'était pas « l'usage ». J'espère, madame la ministre, que vous jugerez que des interpellations en séance publique peuvent relever de « l'usage Face au désengagement d'Engie, pourquoi l'État actionnaire n'a-t-il pas anticipé le besoin de recomposition de l'actionnariat de Suez ? De deux choses l'une : si l'Agence des participations de l'État, prise de court par les turbulences de la crise sanitaire, n'a pas pu mener à bien cette recomposition, il faut le reconnaître. il vous faut assumer le sens de la stratégie consistant à « jouer la montre » qui, faute d'entente entre les parties, était vouée à l'échec. Quand deux des trois acteurs- Veolia et Engie -ont tout intérêt à aller vite, ce n'est pas, à mon sens, une position de neutralité. Le troisième et dernier point de mon sur les conditionnalités. Le Gouvernement entend privilégier autant que possible une intervention directe en fonds propres et non en instruments de dette, assimilables à des fonds propres. L'objectif est clair : en contrepartie de son investissement, l'État veut être en mesure d'exercer une capacité d'influence sur la marche de l'entreprise. Pourquoi, en ce cas, ne pas aller jusqu'au bout de la logique ? Dès lors que l'État entend exercer une capacité d'influence sur la marche de l'entreprise, les conditionnalités se justifient plus que pour tout autre type de soutien public. le mécanisme en vigueur en la matière me semble bien trop timide : comment parler d'« engagements » alors que rien ne vient sanctionner leur Laissez-moi vous faire part de ma conviction. Compte tenu de l'effort massif consenti par la puissance publique, je considère que ce soutien doit être assorti d'exigences. Pour toutes ces raisons, la commission des finances n'a pas adopté les crédits du compte

madame la ministre, mes chers collègues, le budget pour 2021 concernant les investissements d'avenir est caractérisé par deux éléments saillants : la poursuite du PIA 3 dans le contexte de la crise sanitaire, et le lancement d'un PIA 4 en en soutien au plan de relance. Je ne m'étendrai pas sur le PIA 3, si ce n'est pour saluer la souplesse dont cet outil a fait montre cette année. En effet, le secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, a mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros pour soutenir financièrement les entreprises en difficulté ou encore renforcer les moyens dévolus à la recherche en santé. Les programmes d'investissements d'avenir (PIA) ont permis d'apporter des réponses concrètes, ciblées et rapides aux défis posés par la crise sanitaire. La capacité de réaction du SGPI et des opérateurs mérite donc d'être saluée. certaines de ces initiatives devraient se poursuivre. Je pense, notamment, à la création d'une enveloppe d'investissement consacrée à la souveraineté technologique, intitulée « French Tech Souveraineté », et dotée de 100 millions d'euros dans le PLF pour

Je tiens à rappeler, en préambule, qu'il avait été décidé de lancer ce programme avant l'émergence de la covid-19. Il va de soi, cependant, que la crise que nous traversons a fait émerger de nouvelles priorités. Le PIA 4 est doté de 20 milliards d'euros et structuré en deux volets, qui répondent à des finalités distinctes. Un premier volet, dit « dirigé », », vise à financer des investissements exceptionnels, à hauteur de 12,5 milliards d'euros. Un second volet, dit « structurel », doit garantir, grâce à des dotations en capital, un financement pérenne aux écosystèmes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation mis en place par le PIA, à hauteur de 7,5 milliards d'euros. Je ne m'étendrai pas sur les modalités de budgétisation et de gouvernance de ce PIA, qui sont sensiblement identiques à celles du PIA 3 et dérogent tout autant aux grands principes budgétaires. Plusieurs aménagements sont néanmoins apportés à cette gouvernance, pour mettre en oeuvre les recommandations du comité de surveillance des investissements d'avenir. L'article 55, rattaché à la mission, détaille ces modifications : il s'agit, notamment, de la création d'un conseil interministériel de l'innovation pour décider des priorités de la politique d'innovation, du renforcement du rôle du comité de surveillance des investissements d'avenir et de la formalisation d'une doctrine d'investissement pour les investissements Ces évolutions sont bienvenues ; elles contribueront à renforcer la cohérence et l'efficacité des investissements d'avenir. Je voudrais enfin relever l'existence de plusieurs pierres d'achoppement dans ce quatrième programme. Le lancement d'un nouveau programme semble augurer d'un nouveau programme semble augurer d'une pérennisation des investissements d'avenir. La prorogation de ces dispositifs dérogatoires aux règles budgétaires n'est pas problématique en tant que telle, tant que le Parlement demeure à même de suivre et de contrôler l'emploi des crédits qui sont votés. Or il me semble que la maquette budgétaire qui nous est présentée risque d'aggraver le déficit de lisibilité dont souffrent les PIA, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, la liste des secteurs stratégiques qui bénéficieront d'un soutien dans le cadre du volet dirigé du PIA n'est pas encore arrêtée. Nous sommes donc appelés à voter des crédits sans savoir à quels secteurs ou filières ils seront destinés. si je comprends pleinement la logique qui sous-tend cette présentation, j'espère que vous nous exposerez dans les mois qui viennent les stratégies d'accélération qui seront retenues. Je regrette, en parallèle, que deux programmes d'investissement d'avenir coexistent au sein de la mission. Le suivi des montants inscrits dans le PIA 3 se révélait déjà particulièrement complexe, avec la double comptabilité induite par le circuit de la dépense, la dispersion des crédits, l'ampleur des redéploiements en cours de gestion ... Avec ce nouveau PIA 4, qui financera les mêmes structures que le PIA, notre tâche risque de devenir encore plus ardue. Pour terminer, je souhaiterais évoquer l'articulation entre les PIA et le plan de relance. En effet, le PIA 4 doit abonder le plan de relance à hauteur de 11 milliards d'euros sur les trois ans à venir. À mes yeux, une clarification s'impose : les PIA constituent non pas un outil de relance, mais d'investissements à long terme afin de renforcer la croissance potentielle. En pratique, le décaissement des crédits du PIA peut être particulièrement long : trois ans après le lancement du PIA 3, si 4,7 milliards d'euros de crédits de paiement ont été consommés, seuls 750 millions d'euros ont été décaissés. Par conséquent, madame la ministre, il me semble très ambitieux de considérer que les 11 milliards d'euros du PIA 4 pourront irriguer à très court terme le tissu économique français. En dépit de ces quelques réserves, je vous propose d'adopter

Notre commission a donc donné, une nouvelle fois, un avis défavorable sur les crédits de ce compte. L'information transmise au Parlement à propos de ce compte est bien trop lacunaire. Les montants sont « notionnels », c'est-à-dire qu'ils n'engagent en rien le Gouvernement et qu'ils ne permettent pas de connaître ses intentions en matière d'évolution du portefeuille. C'est ainsi par la presse, en dépit de nos questions, que nous avons appris, il y a dix jours, que des négociations sont en cours pour de nouveau renforcer les fonds propres d'Air France-KLM. En outre, cet outil retrace de plus en plus des opérations qui n'ont pas de lien avec l'État actionnaire. La quasi-totalité des recettes de 2021 inscrites sur ce compte seront ainsi des versements budgétaires. Il me semble pourtant que nous pourrions trouver des solutions plus appropriées pour la bonne information du Parlement. Aucun pan de l'action du Gouvernement ne saurait échapper à son contrôle : il s'agit là de l'une de ses missions Ensuite, la stratégie même de l'État est source d'interrogations : il semble de plus en plus devenir actionnaire et de moins en moins stratège. Au fil de ses désengagements successifs, souvent pour des raisons budgétaires, l'État a perdu de son influence et de sa capacité à peser sur certaines décisions pourtant fondamentales pour notre souveraineté économique ou industrielle. Le fait qu'il n'ait pas pu, pas su ou pas voulu défendre ses intérêts dans l'épisode Véolia-Suez découle directement de la baisse continue de sa participation dans Engie. De même, l'accord de cession des Chantiers de l'Atlantique à Fincantieri, toujours sur la table, illustre le privilège accordé au désengagement à court terme, alors même que cet accord est loin de présenter des garanties suffisantes, comme l'a montré un récent rapport du Sénat. Le risque est en effet important que l'acquéreur finisse par rapatrier une partie de sa production en Italie et qu'il procède à des transferts de technologie vers la Chine. Ces constats sont particulièrement alarmants alarmants pour la reconquête de notre souveraineté économique et industrielle, qui nécessite au contraire un État doté d'une vision stratégique à long terme. Enfin, la vraie nature du Fonds pour l'innovation et l'industrie apparaît de plus en plus clairement.

baisse de son rendement. Voilà, mes chers collègues, les raisons qui conduisent la commission des affaires économiques à donner un avis très défavorable à l'approbation de ce compte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la dette est une bombe à retardement pour les Français. La France n'est pas classée parmi les pays frugaux, bien au contraire ! À cet égard, je me permets une observation : le montant de la dette atteindra 120 % de notre PIB, soit plus de 2 600 milliards d'euros,

Nous sommes systématiquement mis devant le fait accompli. Cette situation valait déjà auparavant, mais la tendance s'est considérablement accélérée du fait de la crise sanitaire.

en responsabilité de leurs convertibilités. Le hiatus est trop grand entre la technique du franc CFA et la façon dont celle-ci est reçue dans les pays d'Afrique qui l'appliquent. C'est la raison pour laquelle je serais favorable à une réforme beaucoup moins cosmétique et beaucoup plus

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits de trois missions distinctes : « Remboursements et dégrèvements », « Engagements financiers de l'État » et « Investissements d'avenir

L'intérêt de cette discussion réside surtout dans le lien entre les engagements du passé et les investissements du futur. Notre dette publique montre en effet combien les décisions que nous avons prises par le passé pèsent sur notre futur. En l'occurrence, l'année 2020 s'est avérée particulièrement lourde de conséquences. En moins d'un an, notre taux d'endettement a bondi de 20 points de PIB. En clair, les décisions que nous avons prises dans le feu de l'action de cette crise pèseront encore longtemps sur nos décisions en matière économique et surtout sur nos finances publiques, qui s'en trouveront durablement dégradées. Un chiffre, parmi les 39 milliards d'euros de la mission « Engagements financiers de l'État », illustre bien cette réaction soudaine : les crédits ouverts sur le programme 114, « Appels en garantie de l'État », ont été multipliés par 26,

alors que notre dette explose, la charge de la dette, elle, diminue. L'annulation de 2 milliards d'euros de crédits trahit, à cet égard, la politique européenne de taux bas qui caractérise le contexte macroéconomique actuel. Mais cela durera-t-il ? Cette baisse en trompe-l'oeil contraste nettement avec l'explosion des besoins de financement, qui sont passés de 220 milliards à 362 milliards d'euros. Cette situation a, en outre, obligé l'État français, pour la première fois de son histoire, à se financer par l'emprunt plus que par l'impôt.

du PIA 4 et de ses 11 milliards de crédits au plan de relance nous laisse espérer que notre pays se donnera les moyens de renouer au plus vite avec une croissance renouvelée et durable de long terme. Les PIA permettent d'accompagner notre pays vers des stratégies d'avenir indispensables, comme l'a dit M. le rapporteur

face à la crise. Cela témoigne du soutien de l'État à l'économie, et nous nous en félicitons. Mais le choix gouvernemental d'en passer par l'emprunt sur les marchés financiers doit être interrogé. Cet argent aurait pu être levé différemment, notamment sur l'épargne surnuméraire issue de la crise.

Tout d'abord, les crédits de la mission « Engagements financiers de l'État » sont d'un montant de 39,2 milliards d'euros en 2021, en hausse de 1,93 % par rapport à 2020. Cette mission représente ainsi la troisième mission du budget général de l'État en crédits de paiement. Deux programmes sur cinq, le programme 117, « Charge de la dette et trésorerie de l'État », d'une part, et le programme 114, « Appels en garantie de l'État », d'autre part, représentent à eux seuls 99 % des crédits. Nous pouvons formuler deux remarques à ce propos. D'une part, la charge de la dette reste maîtrisée, et ce malgré un contexte exceptionnel : la hausse de l'endettement public de près de 20 points de PIB et un besoin de financement important.

D'autre part, les garanties octroyées par l'État constituent le principal facteur de hausse des crédits de la mission. Ce montant tout à fait exceptionnel, multiplié par 26 pour 2021, vise à faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Sur la mission « Investissements d'avenir », le budget pour 2021 est caractérisé par deux éléments notables : la poursuite du programme des investissements d'avenir dans le contexte de crise sanitaire, et le lancement d'un PIA 4, en soutien du plan de relance. participera à hauteur de 11 milliards d'euros sur trois ans au plan de relance, dont 6,5 milliards d'euros pour financer des investissements stratégiques et 4,5 milliards d'euros pour les écosystèmes d'innovation. Au travers du PIA, il sera question de cibler certains secteurs, marchés et technologies qui sont considérés comme prioritaires pour la résilience et la souveraineté de notre économie, ainsi que pour la transition écologique et énergétique. Enfin, le budget pour 2021 relatif aux remboursements et dégrèvements constitue une rupture depuis 2010, puisqu'une baisse très nette de 15 milliards d'euros portera les crédits de la mission à 126 milliards d'euros. Cette baisse s'explique par plusieurs facteurs, et tout d'abord, en partie, par l'évolution spontanée des recettes. Du fait de la crise économique, les entreprises ont pu obtenir le remboursement accéléré de leur crédit d'impôt de TVA et de certains crédits Ensuite, cette baisse peut s'expliquer par l'augmentation du coût des contentieux fiscaux pour près de 4 milliards d'euros. Enfin, et pour la première fois depuis 2013, la dépense s'inscrit en nette diminution et recule de 26 milliards d'euros. En matière d'impôts d'État, cette évolution s'explique par le contrecoup des fortes hausses enregistrées en 2020, lesquelles ne se renouvelleront pas en 2021. En matière d'impôts locaux, la suppression du dégrèvement de taxe d'habitation pour 80 % des ménages fera diminuer la dépense de 14,2 milliards d'euros, tandis que la réforme des impôts de production conduira à une baisse de 2,1 milliards d'euros. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe RDPI votera les crédits de ces trois missions discutées simultanément.

madame la ministre, mes chers collègues, comme chaque année, l'établissement de l'ordre du jour du PLF nous conduit à examiner en une seule et même discussion trois missions et quatre comptes financiers et spéciaux, qui touchent à des sujets pourtant assez différents,

une charge de la dette maîtrisée dans la mission « Engagements financiers de l'État » ; la dernière phase du PIA 3 et le début d'un PIA 4 dans la mission « Investissements d'avenir La mission « Remboursements et dégrèvements », au libellé certes peu engageant, reflète néanmoins la gestion du recouvrement des impôts par l'administration fiscale. À 126 milliards d'euros contre 141 milliards l'an dernier, elle concerne toujours principalement les impôts d'État, en particulier la TVA et l'impôt sur le revenu. Je rappellerai à ce titre l'initiative, prise par le groupe du RDSE et notre ancien collègue Yvon Collin, d'un débat sur la fraude à la TVA transfrontalière, qui s'était tenu l'an dernier sur ce sujet majeur et pourtant mal connu. ce qui concerne la mission « Engagements financiers de l'État », la charge de la dette, portée par le programme 117, reste sous le seuil symbolique des 40 milliards d'euros, et continue même de décroître. C'est une bonne nouvelle à court terme, bien qu'il s'agisse toujours- ne l'oublions pas -du troisième poste budgétaire de l'État, après l'enseignement et la défense Le risque de taux sera remplacé petit à petit par un risque de volume de la dette, désormais colossale. Les atouts de la France en la matière restent les mêmes : liquidité et maturité raisonnable de sa dette publique. La diversité des détenteurs lui permet de ne pas dépendre d'un seul ou de quelques-uns qui feraient peser sur notre pays un risque pour sa souveraineté. Rappelons néanmoins que la France est, avec le Royaume-Uni, le seul pays au monde à ne pas avoir fait défaut sur sa dette depuis plus de deux siècles. Le désendettement de la Grèce reste un sujet d'actualité, alors que nous reversons à nos partenaires hellènes les intérêts perçus sur les emprunts qu'ils ont dû contracter. Il faut saluer les importants efforts effectués par ce pays depuis 2010 pour redresser ses finances publiques vrai, un coût social élevé. Aussi, nous devons nous assurer que les intérêts perçus sont bien remboursés intégralement à l'État grec, car il serait incompréhensible de réaliser des profits sur ce compte. J'en viens maintenant à la mission « Investissements d'avenir », qui a pour objet principal le soutien à la recherche, domaine crucial pour l'avenir de notre pays. La diminution du PIA 3 est en trompe-l'oeil puisque les investissements d'avenir vont continuer sous une quatrième forme, portée par l'article 55 rattaché. On serait tenté d'y voir une sorte de continuité, malgré la rupture importante que nous avons vécue cette année en matière de dépenses publiques. Comment le Gouvernement compte-t-il articuler la montée en charge de ce nouveau PIA et les crédits du plan de relance dont nous allons terminer l'examen ce soir ? Après ces quelques remarques nécessairement courtes, je précise que le groupe du RDSE devrait approuver les crédits de ces différentes missions.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « c'est une chose redoutable que les propos du peuple animé par le ressentiment, et l'on paye toujours sa dette à la malédiction populaire », disait l'Agamemnon d'Eschyle. Nos concitoyennes et nos concitoyens sont attentifs aux dépenses, aux politiques, mais également aux modalités de financement. La dette ? L'impôt ? Les taxes ? Pour qui ? Combien ? de la première partie du projet de loi de finances, ce n'est pas faute d'avoir proposé de taxer ceux qui bénéficiaient de la crise et de ceux dont le revenu a augmenté, qu'il s'agisse des grandes entreprises, des géants du numérique ou des 1 % de nos Ce n'est donc pas une fatalité, c'est un choix politique délibéré et assumé : vous n'augmenterez pas les impôts des plus riches. L'explosion de la dette publique à 120 % aujourd'hui n'était pas inéluctable ; vous l'assumerez. La phrase devenue célèbre du Président Macron, selon laquelle « il n'y a pas d'argent magique », nous surprend. Notre pays émet des titres à moyen terme à un taux d'intérêt de 0,2 %, et à court terme à des taux négatifs. On nous paye donc pour financer nos investissements et nos services publics. Je ne sais pas si l'argent est magique, mais la planche à billets n'a jamais produit autant de milliards ! Le poids des intérêts de la dette, il faut que les Français le sachent, diminue tous les ans. L'année dernière, cette dépense s'élevait à 8,63 % des dépenses totales de l'État. Entre 2019 et 2021, la charge de la dette a diminué de 5 milliards d'euros et elle ne représente plus que 37 milliards d'euros chaque année. C'est bien peu au regard du volume de dette, qui devrait atteindre 2 500 milliards d'euros en 2021. En outre, la BCE a pris en charge ce surplus d'émissions dû à la crise sanitaire. Pourquoi nous parler d'un cantonnement de la dette covid ? Elle a été rachetée en totalité par la BCE Nous sommes prévenus : après la crise, ce sera « réforme structurelle » et « réduction des dépenses publiques ». Traduction : réforme des retraites et politique austéritaire ! Encore une fois aveuglés par votre libéralisme dogmatique,

pourrait augmenter le PIB de 2,7 %, l'investissement privé de 10 % et, surtout, créer entre 20 et 33 millions d'emplois, directement et indirectement. » Investir par la dette ? Oui, mais dans quoi ? Mes chers collègues, il faut renforcer nos services publics ! Prenons l'exemple de l'énergie. C'est un bien commun, et un service public national au croisement des enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité et de souveraineté industrielle. Votre stratégie, madame la ministre, consiste aujourd'hui en un désengagement progressif de l'État dans deux entreprises, et surtout en la désintégration de deux entités, EDF avec le projet Hercule et Engie avec un projet de scission de l'entreprise en deux. En voici les conséquences : hausse des tarifs pour les usagers ; détérioration des conditions de travail et perte de statut pour les salariés ; perte

totalement. Il est impératif de changer le statut de ces deux entreprises. Il faut retrouver un véritable service aux usagers, grâce à la création d'un établissement public. Le marché nous a montré ce qu'il engendrait retrouvons un monopole d'État pour l'énergie afin de garantir un service de qualité pour tous, indépendamment des intérêts financiers. Se chauffer, se laver, se nourrir, cela ne saurait être mis à mal par la distribution de dividendes ! La relance doit être l'occasion de rappeler nos fondamentaux, et notamment l'investissement public. La dette n'est pas le problème, mais bien la solution. Cessez de vouloir nous apitoyer en évoquant son poids pour les générations futures ! C'est en agissant pour celles qui vivent aujourd'hui

en 2020, les remboursements et dégrèvements devraient atteindre 152 milliards d'euros. C'est en 2016 qu'ils ont dépassé la barre symbolique des 100 milliards d'euros. Depuis le début des années 2000, l'augmentation est ainsi de 5 % par an en moyenne. Avec la crise sanitaire, et donc incidemment la crise économique, ce budget pour 2021 constitue une rupture puisque la dépense devrait fortement diminuer et s'établir à 126 milliards d'euros, pour la première fois depuis 2013. Ce recul serait de 26 milliards d'euros. En matière d'impôts locaux, la suppression du dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80 % des ménages fera diminuer la dépense de 14,2 milliards d'euros, tandis que la réforme des impôts de production conduira à une baisse de 2,1 milliards d'euros. Il est également à noter que les années 2020 et 2021 devraient aboutir à la clôture budgétaire de procédures contentieuses longues et très coûteuses pour l'État. En 2020, les dépenses au titre des contentieux de série atteindront ainsi près de 4 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 2,6 milliards d'euros au titre d'un contentieux exceptionnel portant sur l'impôt sur les sociétés. Sur proposition de ma collègue députée Christine Pires Beaune, l'Assemblée nationale a adopté l'année dernière un amendement tendant à demander au Gouvernement de publier les informations relatives aux « règlements d'ensemble ». Je note que ce processus permet désormais à l'administration fiscale de négocier les droits et les pénalités dus par un contribuable faisant l'objet d'un contrôle fiscal. Un fait, toutefois, suscite une interrogation : ce processus n'est pas encadré par les textes et, à l'inverse de la transaction, il n'empêche pas l'action contentieuse ultérieure. L'administration y a recours lorsque le quantum des rectifications est difficile à établir ou lorsqu'il existe un fort aléa juridique. Néanmoins, grâce à ce processus, ce sont près de 1,6 milliard d'euros de modérations qui ont été consenties, dont 1,1 milliard d'euros portant sur les droits ; près du tiers concerne une seule opération. Ce processus peut s'entendre, car il revêt un caractère relativement efficient en termes de retour de l'impôt. Toutefois, eu égard aux enjeux qui lui sont liés et en raison de ses implications du point de vue de l'égalité de traitement entre les contribuables, il paraît primordial de connaître précisément le mode opératoire de ce processus, ainsi que la manière dont il opère. Une traduction législative claire et précise en matière de règlements d'ensemble me paraît ainsi nécessaire.

deux nouveaux programmes sont créés dans le cadre du plan de relance, abondés à hauteur de 16,563 milliards d'euros. On note à cet égard une divergence, liée sans doute à la pluriannualité, par rapport aux annonces gouvernementales.

En tout cas, c'est très clairement ce qui s'est passé pour la fin de l'exécution du PIA 3, ainsi qu'en atteste de manière incontestable le « bleu » budgétaire présenté par le Gouvernement. Pourtant, nous passer de ces crédits d'investissement me paraît une grave erreur, dans le contexte de crise économique que nous traversons, qui rend nécessaire une relance économique forte. Avec la perte en cascade de nos industries, couplée à la tertiarisation de notre société, la France va devoir s'adapter et innover pour rayonner encore dans le monde. En particulier, nous devons nous tourner vers les secteurs d'innovation non délocalisables, qui sont vecteurs d'un savoir-faire bien français.

282 milliards d'euros. Ensuite, le programme 114, « Appels en garantie de l'État », dont les crédits sont multipliés par 26 pour atteindre 2,5

passages de votre rapport. Ainsi, nous ne pensons pas que les montants des restitutions d'impôt aux entreprises témoignent du caractère vicié des fondements de l'Union européenne. Non, nous ne pensons pas non plus que l'Union européenne grève les finances de l'État de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour favoriser la circulation des capitaux et l'égalité de traitement entre les entreprises européennes. Non, nous ne pensons pas davantage que l'Union européenne joue le rôle de cheval de Troie du néolibéralisme. Nous considérons également que les critiques qu'il formule sur les remboursements aux entreprises au titre du crédit d'impôt recherche (CIR) sont quelque peu exagérées

5 %. Nous pensons plutôt que le CIR constitue une aide à l'innovation et doit être préservé pour soutenir l'effort de recherche de notre pays. Je conclurai sur cette mission en posant une question au Gouvernement,

Dans un arrêt du 3 décembre 2018, le Conseil d'État a fixé les règles du contentieux. Puis, en juillet 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que la CSPE pouvait être remboursée partiellement, à proportion de la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale.

Si, demain, la BCE doit revoir sa stratégie d'intervention, notamment pour satisfaire la cour constitutionnelle de Karlsruhe, la Banque de France sera limitée dans ses capacités d'intervention sur le marché secondaire, en sorte que la dette nationale sera beaucoup plus sensible aux exigences des marchés.

part, l'État a utilisé un dispositif assez intéressant à court terme : les primes d'émission sur des souches anciennes. Aujourd'hui, les investisseurs nous donnent de l'argent pour bénéficier de ces souches anciennes. Mais la conséquence directe est que nous allons devoir rembourser plus vite et à un coût plus élevé.

Pouvez-vous nous en dire plus ? Doit-on en déduire un probable cantonnement de l'endettement public, avec la mise en place de recettes spécifiquement destinées à l'amortissement

ont permis de lancer les travaux méthodologiques d'évaluation de la fraude, articulés autour de trois axes : la poursuite des travaux engagés par l'Insee sur la TVA pour déboucher sur des estimations annuelles ; la définition d'une méthode d'évaluation en ce qui concerne les autres impôts, notamment l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu

je tiens à répondre aussi aux préoccupations que vous avez exprimées sur le risque de non-compensation pour les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme des impôts de production. Les compensations prévues par le projet du Gouvernement sont intégrales territorialisées ; pour les régions, elles permettent de substituer à une ressource volatile, la CVAE, une ressource plus stable et plus dynamique.

Par ailleurs, la crise a entraîné un mouvement d'aversion pour le risque favorable au marché obligataire : les taux d'intérêt sur la dette française sont proches des plus bas niveaux historiques. Il est d'ailleurs assez probable que l'épargne

Sur le plus long terme, une hausse des taux d'intérêt est déjà intégrée à la programmation budgétaire du Gouvernement, en cohérence avec un scénario pluriannuel de raffermissement des conditions macroéconomiques. Ainsi, le projet de loi de finances se fonde sur l'hypothèse que le taux à dix ans sera de 0,70 % à

le Gouvernement est soumis à une double obligation : celle d'information et de transparence à l'égard du Parlement et celle de gérer au mieux les deniers publics qui lui sont confiés, donc de défendre les intérêts du contribuable, ce qui suppose de ne pas révéler ses intentions aux marchés.

». Monsieur Lurel, ces versements seront échelonnés : ils interviendront au fur et à mesure des besoins exprimés par l'Agence des participations de l'État et les entreprises concernées en vue de la réalisation d'opérations de crise visant à soutenir, au moyen de fonds propres, de quasi-fonds propres et de titres de créance, des entreprises stratégiques particulièrement fragilisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Si la crise a fragilisé le portefeuille de l'Agence des participations de l'État, elle ne remet pas en cause notre vision de l'État stratège. La structure financière des sociétés du portefeuille de l'agence s'est sensiblement dégradée, entraînant des fragilités qui pourraient perdurer. L'État a su mettre en place et mobiliser des outils de soutien immédiat à la trésorerie des entreprises. Il va désormais intervenir pour renforcer les fonds propres ou les quasi-fonds propres des entreprises stratégiques durablement fragilisées par la crise. C'est l'objet du travail conduit par l'Agence des participations de l'État dès la première vague de la crise sanitaire, en mars et avril en identifiant les entreprises françaises stratégiques les plus vulnérables et en quantifiant les besoins potentiels en renforts de fonds propres. Nouvelle génération d'investissements d'avenir, le PIA 4 permettra d'accélérer l'innovation et la transformation de notre économie.

au côté de partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. Ses investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures sélectives ouvertes et des principes de cofinancement ou de retour sur investissement pour l'État. Dans un contexte où le soutien à l'innovation est plus que jamais nécessaire, nous lançons un quatrième programme d'investissements d'avenir. Massif, il vise trois grandes finalités, désormais inscrites dans sa doctrine : la croissance potentielle, la transition énergétique et écologique et la résilience de nos organisations et de notre économie, qui conditionne notre souveraineté. Ces trois finalités traduisent les priorités et l'ambition du Gouvernement pour la transformation de notre pays sur le long terme. Doté de 20 milliards d'euros, le PIA 4 sera mis en oeuvre, comme l'a expliqué M. Bizet,

un volet structurel de 7,5 milliards d'euros garantira un financement pérenne et prévisible aux écosystèmes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, dont le financement est en grande partie assuré par des dotations en capital produisant, à terme, des revenus réguliers et récurrents.

traduit l'effort de rationalisation des instruments de financement que nous opérons dans cette loi de finances. De plus, nous proposons d'étendre les missions du comité de surveillance des investissements d'avenir, où siègent huit parlementaires, pour mieux vous associer aux grandes orientations d'investissement. C'est une réponse à l'une de vos demandes. ce quatrième PIA comportera une dimension territoriale amplifiée, permettant d'assurer le déploiement des innovations en les adaptant aux réalités des territoires. Très bien ! Les partenariats seront renforcés avec les grands acteurs des territoires, tandis que l'enveloppe de la tranche régionalisée sera doublée, passant de 250 à 500 millions d'euros ; le couple préfet-président de région se verra renforcé dans sa capacité de pilotage. Enfin, le PIA 4

alors que les budgets d'innovation et de recherche et développement pourraient être sacrifiés en période de crise, l'objectif du PIA est de mobiliser des moyens exceptionnels pour ne pas brider l'élan des chercheurs et des entrepreneurs français.

Conformément à la recommandation du comité de surveillance, nous répondons à une demande légitime formulée de longue date par le Parlement en vous proposant d'inscrire dans la loi la doctrine d'investissement du PIA. Cette doctrine, ainsi que la nouvelle gouvernance que nous mettons en place

Le présent amendement ouvre des crédits supplémentaires en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » à hauteur de 696 millions d'euros. Ces crédits correspondent

On peut élaborer des théories ou entendre des choses, mais la réalité, c'est que les entreprises sont contrôlées, particulièrement quand

La crise économique que nous traversons ne justifie pas d'abandonner les grands objectifs qui sont les nôtres, mais également les vôtres, madame la ministre, ainsi que ceux de votre gouvernement en matière d'égalité professionnelle, bien au contraire. Or, vous le savez, madame la ministre, deux tiers des travailleuses indépendantes et des femmes entrepreneurs n'ont maintenu, au mieux, que 20 % de leur activité pendant le confinement, et 54 % considèrent que leur entreprise est aujourd'hui en situation de risque élevé de dépôt de bilan. Cette situation partagée par un nombre important d'entrepreneurs est rendue plus difficile encore pour les femmes en raison des charges qui pèsent sur elles, mais également des difficultés qu'elles rencontrent à se faire financer : 44 % d'entre elles estiment que les échecs de création d'entreprises s'expliquent par le manque de financement, le taux de rejet des crédits demandés par les créatrices d'entreprises étant supérieur

moins de fonds que les start-up créées par les hommes. Ces injustices doivent cesser. Or l'expérience montre que dans tous les domaines, les avancées sur cette question ne se font que lorsque la loi prévoit des mesures contraignantes.

Mme Martine Filleul. Depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, chaque année, avant le 1 mars, les entreprises d'au moins cinquante salariés doivent calculer et publier sur leur site internet leur index de l'égalité salariale Or la ministre du travail a indiqué que 17 000 entreprises n'avaient toujours pas publié leur index. Il est inacceptable, en 2020, que ces inégalités salariales subsistent et que les entreprises ne soient pas mises devant leurs obligations.

madame la ministre,

rapporteure spéciale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la mission « Économie » porte un ensemble de dispositifs en faveur des entreprises, notamment les PME, dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et de l'industrie. Elle porte aussi les crédits des administrations, autorités administratives indépendantes et opérateurs chargés de la mise en oeuvre de ces politiques. Cette année, la mission « Plan de relance » concentre l'ensemble des crédits nouveaux en faveur des entreprises,

du déblocage progressif des crédits de paiement affectés au plan France Très haut débit. En dehors de ces deux mesures, les crédits permanents de la mission sont globalement en baisse et leur réduction à périmètre constant se poursuit. constant se poursuit. Des mouvements de crédits importants ont été opérés sur la mission au cours de cette année. Une nouvelle action dédiée aux mesures exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire a été créée pour couvrir 860 millions d'euros de dépenses urgentes. Elle a porté les crédits de plusieurs mesures d'urgence, comme l'achat de masques à usage non sanitaire et les dispositifs d'aide exceptionnelle au secteur automobile, automobile, aux centres équestres, aux poneys clubs, aux cirques avec animaux, aux parcs zoologiques, aux aquariums ou encore aux refuges. Cette action n'étant pas dotée de crédits pour 2021, nous nous interrogeons, madame la ministre, sur l'avenir de ces dispositifs de soutien, alors même que la deuxième vague de l'épidémie produit des effets délétères pour ces secteurs. Au niveau de la mission, les moyens accordés aux différents dispositifs d'intervention seront en nette diminution pour 2021. Sur le programme 134, une fois exclue la compensation carbone, les crédits alloués aux autres interventions sont passés de 350,2 millions d'euros en 2017 à 165,3 millions en 2021, soit une diminution de 53 %.

portent sur des secteurs très divers, allant de la petite industrie aux métiers d'arts, en passant par les commerces de centre-ville, les services à la personne ou encore les jeunes PME innovantes. Les coups de rabot successifs ne permettent pas de dégager d'orientation politique durable pour la mission « Économie ». Sur le long terme, il faut prévoir un réel désengagement de l'État qui laissera les territoires

ne remettent pas en cause cette logique globale de désengagement. Une fois cette mission arrivée à son terme, l'ensemble des dispositifs d'intervention de l'État en faveur des entreprises risque de disparaître définitivement, puisque les crédits d'intervention du programme 134 continuent de fondre.

Dans le contexte de crise sanitaire et de confinement, les chantiers de déploiement ont pris du retard, ce qui a engendré d'importants surcoûts sur l'ensemble du territoire. Même si nous saluons les efforts réalisés par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, nous considérons que le compte n'y est pas et qu'un effort supplémentaire devra être consenti pour atteindre l'objectif

Dans le contexte de la crise actuelle, nous ne pouvons que saluer la diminution des réductions d'effectifs que nous constatons pour 2021. La pression diminue en particulier sur les administrations du programme 134, la baisse des effectifs passant de 155 suppressions en 2020 à seulement 22 en 2021. Tout d'abord, la réduction des effectifs de la direction générale des entreprises (DGE) devrait être moindre, avec une baisse de 19 équivalents temps plein (ETP) en 2021. Ces derniers mois, les services déconcentrés ont été particulièrement mobilisés, de sorte que la priorité est à la gestion de crise la finalisation du projet de services économiques de l'État en région a été retardée à 2022. L'activité des services doit pouvoir continuer à se focaliser sur l'accompagnement des entreprises en difficulté, ainsi que sur les filières stratégiques et l'innovation. l'innovation. La réduction des effectifs de la direction générale du Trésor se poursuivra en 2021 à un rythme moins soutenu qu'auparavant, avec la suppression de 13 ETP. La rationalisation du réseau a été particulièrement forte au cours des dernières années,

Poste bénéficie, reviennent aux commissions départementales de la présence postale territoriale et au financement des points de contact éligibles. La Poste garantit l'accessibilité de services indispensables pour nombre de nos concitoyens. Je pense en particulier à l'accès au compte et à l'accessibilité numérique.

La sinistralité envisagée avant la mise en oeuvre de nouvelles restrictions pour faire face à la deuxième vague épidémique impliquait un coût global du dispositif de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros, soit un niveau relativement limité au regard des apports du dispositif en termes de soutien aux entreprises. La deuxième vague de l'épidémie et les nouvelles restrictions pourraient cependant faire évoluer ce coût de façon très significative. Le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers et à des organismes privés » comprend les crédits de deux dispositifs qui permettent également de pallier les difficultés de financement des entreprises. Il s'agit, d'une part, du fonds de développement économique et social (FDES), d'autre part, des avances remboursables et prêts bonifiés gérés par la direction générale des entreprises.

Les deux dispositifs ont permis d'octroyer un nombre assez limité de prêts. En effet, à peine plus de 20 % du milliard d'euros prévu pour 2020 a été consommé, de sorte que l'intégralité des crédits sera reportée en 2021, avec une ouverture de crédits complémentaire de 75 millions d'euros.

D'après les informations transmises, une soixantaine de dossiers resterait en instance. Pour conclure, je souhaite aborder la question du concours de l'État au financement des fonds de garantie de Bpifrance. En effet, depuis plusieurs années, Mme Espagnac et mon prédécesseur, Bernard Lalande, déplorent l'absence de budgétisation des crédits dédiés aux fonds de garantie, qui résultent de redéploiements de crédits ou de recyclages internes à Bpifrance. Ces débudgétisations sont en contradiction avec le principe d'universalité budgétaire et nuisent à la sincérité des comptes publics. De plus, pour 2021, des crédits dédiés à ces garanties classiques ont été rangés au sein du plan de relance, alors qu'ils auraient dû être retracés dans le programme 134.

mes chers collègues, mon propos sera essentiellement centré sur les crédits qui concernent le volet « Commerce et artisanat ». Si le plan de relance dédié à ces secteurs regroupe environ 200 millions d'euros de crédits, la mission « Économie », quant à elle, n'en retrace quasiment plus aucun. C'est pourquoi la commission des affaires économiques a adopté quatre amendements. Le premier concerne le Fisac, fonds qu'il ne nous semble pas raisonnable de supprimer, alors même que les autres dispositifs censés le remplacer ne sont pas encore suffisamment opérationnels.

Le troisième amendement concerne l'initiative France Num, devenue la pierre angulaire de la politique publique de numérisation des PME. Bien qu'utile, l'initiative souffre d'une notoriété insuffisante et d'une absence totale de suivi de ses actions et de mesure de leur efficacité. Il nous paraît essentiel, à un moment où la transition numérique semble enfin considérée comme primordiale, de financer une vaste campagne de communication qui ne soit pas ciblée sur les entrepreneurs déjà familiers du sujet, mais au contraire sur tous ceux qui en sont éloignés. La commission a donc adopté un amendement qui tend à augmenter de 5 millions d'euros la dotation de France Num, dans l'objectif de financer également la mise en oeuvre d'un dispositif de suivi des actions de numérisation mises en place grâce à son entremise.

aux crédits, nous vous présenterons un amendement, déjà adopté par le Sénat lors de l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative, mais rejeté par l'Assemblée nationale, tendant à créer un crédit d'impôt à la numérisation et à l'équipement.

Depuis plusieurs années, le Sénat plaide pour un cap clair et des financements conséquents pour développer les réseaux d'initiative publique sur tous les territoires. L'enjeu d'inclusion numérique est bien connu et son caractère essentiel a été ravivé par les confinements successifs.

Le Gouvernement recycle des crédits qui ne sont pas nouveaux, mais ils permettent de mobiliser un total de 550 millions d'euros. Il était temps, madame la ministre, car nous sommes malheureusement toujours les bons derniers de l'Union européenne en matière de très ! Une étape a donc été franchie, en ce qui concerne le soutien aux territoires. Il conviendra à présent de nous assurer que le cahier des charges du plan France Très haut débit permette de financer tous les raccordements, y compris les plus longs et les plus complexes.

Ces missions sont pourtant essentielles, et la crise de ces derniers mois l'a encore prouvé. Dans ce budget, madame la ministre, vous proposez comme seule réponse de diminuer la compensation du service de transport et de distribution de la presse, à moins de 90 millions d'euros. Quand on connaît l'équivalent dont dispose La Poste belge, à savoir 170 millions d'euros, on se demande comment La Poste française pourrait poursuivre une mission de qualité sur un territoire vingt fois plus grand et avec moitié moins d'argent

Nous avions cru comprendre jusqu'alors que c'était une solution acceptable pour le Gouvernement, mais il semblerait que la question ne soit pas encore tranchée et qu'elle reste suspendue à l'arbitrage du Premier ministre. Nous espérons donc, madame la ministre, que vous pourrez nous annoncer une bonne nouvelle, après plusieurs semaines de débat, et

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le choc économique que nous subissons depuis mars a eu pour conséquence d'exacerber les faiblesses structurelles de notre industrie à au moins quatre niveaux. l'endettement s'est accru de 13 % et, en septembre dernier, l'encours total de dette de l'industrie était proche de 150 milliards d'euros, ce qui est d'autant plus problématique que les entreprises industrielles françaises sont faibles en fonds propres. Ensuite, l'investissement a chuté de 14 % par rapport à 2019, alors que notre outil industriel a dix-neuf ans d'âge moyen. Il est deux fois plus ancien qu'en Allemagne, et bien moins robotisé et numérisé.

La crise a aussi révélé l'importante dépendance de notre économie à certains grands secteurs exportateurs comme l'aéronautique et, dans une moindre mesure, l'automobile. Au-delà du seul déficit de notre commerce extérieur, le risque est que nous perdions durablement des parts de marchés à l'international.

d'abord, un soutien plus conséquent à la demande sera nécessaire, car la crise qui se profile fera des dégâts dans l'ensemble de l'industrie. Plusieurs leviers existent, dont le soutien à des secteurs oubliés du plan de relance, comme la construction neuve, qui encourage en particulier la production métallurgique. La commande publique en est un autre, mais encore faudrait-il que les collectivités qui représentent 60 % de l'investissement public disposent des ressources nécessaires.

longtemps attendue de penser une politique industrielle souveraine, ambitieuse et réaliste, qui utilise tous les leviers de transformation de notre industrie. Les orientations stratégiques de la réindustrialisation du pays devraient faire l'objet d'une implication directe du Parlement, en concertation avec les filières et les régions. et les régions. Si le plan de relance identifie bien les enjeux de long terme, il doit être renforcé à court terme pour pallier une crise de la demande et mieux anticiper le problème de l'endettement. La commission des affaires économiques a émis un avis favorable à l'adoption

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la question de la juste intervention publique dans la sphère économique nourrit d'intenses débats depuis plusieurs siècles. En cette année 2020, et dans les circonstances que nous connaissons, La mission « Économie » se compose de quatre programmes principalement orientés vers l'accompagnement des entreprises, notamment pour la transition numérique de l'artisanat et des petites entreprises. L'enjeu est essentiel dans le contexte actuel.

Si nous saluons les efforts financiers tout à fait nécessaires engagés depuis le début de la crise pour aider les entreprises, des réponses plus fortes doivent être apportées pour accompagner le tissu économique dans son ensemble. Concernant les crédits de la mission, la hausse que nous constatons cette année résulte de la nette augmentation des crédits du dispositif de compensation carbone des sites électro-intensifs et du programme 343, « Plan France Très haut débit »- les crédits À ce sujet, il nous paraît nécessaire de donner la priorité à la couverture des zones blanches demeurant en France avant d'achever la couverture en très haut débit. Nous regrettons par ailleurs le manque de lisibilité globale de cette mission du fait du plan de relance qui fait l'objet d'une mission spécifique, ce qui, si cela se justifie d'un point de vue opérationnel,

l'unanimité ce soir -, voulue par le Gouvernement, n'a pas de sens. La crise actuelle affecte en premier lieu l'artisanat et le commerce. Il est indispensable de disposer de crédits d'intervention, afin de maintenir ces activités dans nos territoires les plus fragiles, notamment ruraux. C'est pourquoi nous soutiendrons les amendements visant à rétablir les crédits du Fisac à hauteur de 30 millions d'euros. Nous regrettons bien entendu l'absence de conditionnalité

Plus largement, nous regrettons l'opposition de ce gouvernement à toutes nos propositions tendant à instaurer des solidarités économiques nouvelles, comme la contribution exceptionnelle sur les géants de la vente en ligne. Mettre fin à la distorsion de concurrence entre le commerce de proximité et le commerce en ligne est un enjeu d'équité et de justice sociale et fiscale- c'est une question qui est au coeur des préoccupations des acteurs du tissu économique local cher à nos concitoyens. Une réflexion de fond doit aujourd'hui être menée en vue d'inventer une fiscalité du commerce répondant aux enjeux écologiques du XXIsiècle et permettant de lutter réellement contre les stratégies d'évitement de l'impôt mises en place par certains géants du numérique. Vous parlez de souveraineté et de relocalisation, mais nous attendons toujours les actes nous assurant de reprendre la maîtrise de notre système productif. Garder le monopole sur nos fleurons nationaux est également essentiel nous attendons le retour d'un État stratège. Utilisons si nécessaire la nationalisation provisoire pour conserver sur le sol français des capacités en matière de production stratégique. Je pense par exemple à Luxfer, dernière unité de production en Europe de bouteilles d'oxygène médical, une entreprise menacée de fermeture définitive.

Si nous ne nous opposons pas à l'ensemble des mesures, nous ne pouvons pas approuver un budget conçu selon une doctrine néolibérale fondée sur la compétitivité des entreprises et la consommation à tout prix, objectifs qui ne répondent pas aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.

de la compétitivité des entreprises et de la résilience économique de la France. Pour la mission « Économie » en tant que telle, les crédits sont en augmentation de près de 14 %. Cette hausse est liée à l'évolution du montant de la compensation carbone accordée à certaines entreprises, d'une part, et au déploiement du plan France Très haut débit au titre du programme 343, d'autre part. En début de mandature, le Président de la République a fixé l'objectif d'une couverture intégrale du territoire national en haut débit d'ici à 2020, et en très haut débit d'ici à 2022. Afin d'y parvenir, le programme d'investissements d'avenir (PIA) piloté par le secrétariat général pour l'investissement représente la première source de financement. À cela viennent s'ajouter plusieurs ressources complémentaires prévues dans ce programme, en soutien aux réseaux d'initiative publique des collectivités. Les projets sont quasi finalisés : leur intervention doit garantir l'utilisation partagée du réseau et respecter le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés. Les crises sanitaire et économique que nous traversons impliquent en effet la sécurisation et la généralisation de la couverture en fibre optique sur l'ensemble du territoire, mais elles nécessitent aussi de prendre en compte la dégradation des conditions financières et le cofinancement des raccordements coûteux pour les sites les plus isolés. En parallèle, saluons l'initiative de former 4 000 médiatrices et médiateurs, afin de lutter contre l'illettrisme et la fracture numériques ; cette politique est d'autant plus nécessaire que la période de confinement a accru l'usage des services numériques pour l'accès à des services essentiels de la vie quotidienne. Les politiques publiques financées par le programme 134 visent, quant à elles, à redynamiser l'environnement économique, en ciblant trois objectifs stratégiques : développer les PME et les entreprises de taille intermédiaire, en renforçant l'offre classique de garantie des prêts de Bpifrance renforcer le soutien à l'international des entreprises à l'export, en particulier grâce au travail de Business France ; enfin, réguler et sécuriser les marchés pour s'assurer du respect des règles de concurrence, ainsi que de la qualité et de la sécurité des produits mis sur le marché.

Enfin, le programme 305 prévoit les moyens de fonctionnement de la direction générale du Trésor. Son action de conception et de mise en oeuvre des politiques économiques et financières visera un objectif essentiel, celui de retrouver dès 2022 un niveau de richesse nationale équivalent à celui d'avant la crise, mais

les différents rapporteurs l'ont déjà mentionné, le projet de loi de finances pour 2021 est profondément marqué par la crise sanitaire, économique et sociale que nous vivons depuis le mois de mars.

Concernant les programmes de cette mission, il y a plusieurs points, sur lesquels j'aimerais revenir. D'abord, j'évoquerai le ralentissement des réductions d'effectifs à la DGCCRF, ainsi qu'à la direction générale des entreprises.

le but n'étant pas de contrôler pour le plaisir de sanctionner, mais bien de protéger nos petites et moyennes entreprises et de faire respecter la législation en matière de transition écologique.

Concernant les différentes aides aux entreprises, il convient de souligner leur nombre et le soutien déterminant qu'elles apportent à l'économie locale. Je pense notamment aux prêts garantis par l'État, gérés par Bpifrance. Au total, un encours de 300 milliards d'euros sera financé, avec une garantie de deux ans de décalage pour le remboursement.

Plus que jamais, nous devons rappeler notre attachement à ce dispositif qui, s'il n'est pas parfait, permet de compenser de nombreux freins à l'installation dans nos territoires ruraux. J'émettrai la même critique que nos collègues rapporteurs sur le manque de visibilité et l'absence de pilotage global des différents mécanismes de soutien à l'activité économique. Sur le soutien aux commerces ruraux, je soutiendrai là encore l'amendement des rapporteurs spéciaux concernant le Fisac. Le souhait de l'enterrer, qui s'accompagne d'une baisse de 80 % des crédits qui lui sont dévolus, est une erreur, d'abord parce que la crise que nous connaissons vient de démontrer l'importance de nos commerces de proximité,

Pour conclure, à l'instar des rapporteurs, nous plaidons pour une plus grande lisibilité, une plus grande coordination des aides à destination des entreprises et pour que l'action publique, au niveau national comme sur nos territoires, soit encore simplifiée.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous déplorons que, dans ce projet de loi de finances pour 2021, les crédits consacrés à l'économie soient éparpillés entre la mission « Économie » et le plan de relance. Malgré l'illisibilité qui en découle, les lacunes sont évidentes le commerce de proximité et l'artisanat représentent 3 millions d'entreprises et 3,5 millions de salariés. Une seule question compte : combien d'entre elles baisseront définitivement le rideau après les deux confinements que nous venons de vivre ? de ces fermetures, combien de personnes auront tout perdu, leur commerce pour les petits patrons, leur travail pour les salariés, mais aussi leur maison et leurs économies pour beaucoup

Vous me répondrez qu'il y a le chômage partiel, le fonds de solidarité et les prêts garantis par l'État, mais le problème, c'est que le Gouvernement est fort avec les faibles et faible avec les puissants. Par exemple, plutôt que de travailler à une réouverture des librairies, vous avez fermé les rayons « culture » des hypermarchés. Pendant ce temps, Amazon et les autres géants du e-commerce ont tranquillement régné pendant entre autres secteurs. Et alors qu'Amazon paie peu d'impôts et participe activement à la fraude fiscale à la TVA de ses revendeurs intracommunautaires, le ministre de l'économie s'est félicité d'avoir fait reculer le Black Friday d'une semaine- la belle affaire ! Amazon s'en est félicité pour en pour en récupérer le mérite et se donner une image vertueuse après un mois de profits au détriment des commerces de proximité. Nous aurions préféré légiférer pour imposer à Amazon une taxe alimentant le fonds de solidarité. Aujourd'hui, les commerces rouvrent : c'est bien, mais c'est insuffisant, car il va leur falloir compenser plusieurs mois de fermeture. Et ce sera pire pour les restaurants, les cafés et leurs personnels, dont les revenus dépendent en partie des pourboires- ils devront attendre le 20 janvier prochain. S'ajoutent à cela les difficultés d'accès au fonds de solidarité malgré quelques avancées, obtenues notamment par le Sénat. Par exemple, pourquoi les gérants salariés en sont-ils encore exclus, alors qu'ils cotisent pour l'ensemble des risques et qu'un patron affilié

partiel avant même le reconfinement de novembre. M. le ministre de l'économie l'a d'ailleurs reconnu sur France Inter cette semaine : « Les salariés font des efforts considérables et la vie est difficile pour eux.

le sursaut économique aussi attendu que souhaité par tous les acteurs politiques et économiques dépendra avant tout de notre capacité à sortir de la crise sanitaire. Avec une chute d'activité de 12 % en novembre contre 31 % en avril, il est difficile de mesurer aujourd'hui la capacité de notre économie à reprendre vite et fort, mais le déconfinement de l'été nous permet d'être un peu plus optimistes. Cependant, cette reprise ne sera réelle que si la casse économique est limitée et si les entreprises sont accompagnées au maximum. Les plans d'urgence et de relance proposés par le Gouvernement constituent des réponses indispensables à la marche de l'économie. On peut se réjouir de leur existence et des mesures qu'ils prévoient. on peut néanmoins regretter la difficulté à lire les crédits consacrés à la relance qui se trouvent à la fois dans la mission « Économie » et dans la mission « Plan de relance », examinée il y a deux jours. La mission « Économie » a d'ailleurs servi d'outil, dès cette année, notamment pour porter les prêts garantis par l'État et les prêts à taux bonifiés. Pour que la reprise soit efficace, il faut qu'elle irrigue tous les territoires, qu'elle touche les populations les plus en difficulté et qu'elle anticipe l'avenir. C'est pourquoi j'aimerais, à ce stade, insister sur quelques points. Tout d'abord, la vitalité des territoires ruraux et la survie de certains centres-bourgs dépendront du dynamisme du commerce de proximité et de l'artisanat.

Nous voterons donc l'amendement proposé par la commission des finances pour rétablir cet outil simple et primordial. Très bien ! Ensuite, préparer l'avenir, c'est déployer le très haut débit sur tout notre territoire.

Les objectifs sont bons, mais pourriez-vous, madame la ministre, faire un point sur les réalisations ? Ne passons pas non plus à côté de la couverture de tout notre territoire parler de la 5G, c'est bien, mais prenons garde de ne pas accentuer la fracture numérique. Aujourd'hui, la précarité se développe. Les plus jeunes habitants des zones rurales sont les plus en difficulté. Enfin, la crise que nous traversons a mis en lumière les difficultés de notre économie mondialisée : problèmes liés aux délocalisations des activités industrielles, manques de compétences, problèmes d'approvisionnement et difficultés d'exportation. La santé et l'alimentation sont devenues des secteurs essentiels : l'État doit définir clairement sa stratégie en la matière pour protéger,

Il y va aussi du développement du commerce extérieur et, donc, de la balance commerciale de la France. Madame la ministre, nous aurions aimé connaître les ambitions du Gouvernement dans ce domaine.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à la suite de l'intervention du Président de la République le mardi 24 novembre et de celle du Premier ministre le jeudi 26, nous connaissons aujourd'hui les premières mesures de déconfinement après la deuxième vague de la pandémie. Si, dans nos territoires, et pour la première fois depuis plusieurs semaines, quelques-uns de nos commerces, de nos ateliers et autres lieux d'activité ont la possibilité d'ouvrir à nouveau, les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de l'année 2020 ne sont pas pour autant surmontées ni résolues. C'est dans ce contexte singulier et particulier que les sénateurs et sénatrices socialistes, écologistes et républicains vous font part de leur analyse et de leurs remarques sur les crédits de la mission « Économie

Mais notons-le, comme elle n'est pas dotée de crédits spécifiques pour l'année 2021, se posera la question de savoir où seront ponctionnées les ressources budgétaires en cas de besoin. Par ailleurs, la mise en oeuvre d'un plan de relance de l'économie doté de 100 milliards d'euros sur deux ans a certes recueilli les faveurs de l'opinion publique, mais il ne faudrait pas que les effets d'annonce brouillent l'action, certes moins médiatique, mais plus pérenne du programme 134 et des autres programmes de la mission.

Leurs besoins sont immédiats, mais doivent aussi trouver des réponses dans la durée. Le projet de budget entérine la réorganisation de la direction générale des entreprises sur nos territoires, avec notamment la création des services économiques de l'État en région et la mise en place de pôles « entreprises, emploi, économie ». Nous n'en contestons pas le principe, mais ces décisions aboutissent néanmoins à une réduction du nombre des fonctionnaires sur le terrain au moment où leur mission de conseil et de soutien est particulièrement nécessaire. Année après année, les

Comme l'ont souligné nos collègues rapporteurs, il faut faire beaucoup plus pour les PME et les ETI, l'artisanat et le commerce dans nos territoires. Ces activités sont le poumon économique de nos régions et sont le plus souvent très riches en emplois. Selon les calculs de nos collègues, l'effort financier de l'État en faveur des commerces et de l'artisanat a diminué de 89 % en dix ans. Il n'est plus véritablement lisible aujourd'hui, car il dans l'action n° 23. Nous considérons que les activités productives, les commerces et les services de proximité doivent être prioritaires. proposé la création d'une contribution exceptionnelle des acteurs économiques ayant perçu des bénéfices accrus en 2020, comme les assureurs et les acteurs du e-commerce. L'objectif était d'en redistribuer le produit aux acteurs économiques qui ont dû fermer ou dont l'activité s'est effondrée. L'économie de proximité doit être identifiée comme une priorité dans le cadre de la relance économique. Des annonces ont été faites en ce sens en juin 2020 avec, comme mesure principale, un renforcement du soutien à la création de foncières de rénovation commerciale. Cela nous semble bienvenu, mais là encore, au-delà de l'effet d'annonce, nous souhaitons qu'une réponse soit véritablement apportée à la dévitalisation commerciale qui frappe nombre de nos communes, avec un ciblage resserré sur les territoires les plus fragiles.

Par ailleurs, la hausse des crédits dédiés au soutien des entreprises- mes collègues rapporteurs l'ont indiqué -concerne essentiellement la compensation carbone ; elle cache en réalité une diminution de 53 % des crédits, hors compensation carbone. Il est indispensable, dans la situation actuelle, de rétablir de façon pérenne ces crédits et d'élaborer une véritable stratégie de pilotage du soutien aux entreprises. Au-delà de ces réserves, les rapporteurs spéciaux proposent des avancées significatives pour soutenir efficacement l'activité de proximité, à savoir le maintien du Fisac et le renforcement de ses moyens, mais aussi une hausse des crédits alloués au plan France Très haut débit. Ils proposent également de garantir le maintien d'une présence postale sur l'ensemble des territoires. Ce sont ces mesures que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain soutient fortement, car elles auront des effets immédiats et visibles pour nos concitoyens, nos commerces et nos artisans. Si ces amendements sont adoptés, mon groupe votera les crédits de la mission. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention s'articulera autour de deux axes. Le premier concerne le numérique et, plus particulièrement, le plan France Très haut débit. L'année dernière, nous avions dû batailler pour faire adopter un amendement tendant à abonder ce plan, amendement rejeté sans autre forme de procès par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

ce qui prouve bien, madame la ministre, que nous avions raison il y a un an de vouloir augmenter les crédits du Fonds pour la société numérique. Notre position n'était en rien « détestable »- votre

C'est d'autant plus vrai que l'État dispose encore de près de 50 millions d'euros de subventions aux opérateurs privés inutilisées dans le cadre du guichet de cohésion numérique des territoires, subventions qu'il convient de flécher à nouveau vers l'achèvement de la couverture FTTH du territoire.

Mais, pour que rien ne vienne entacher ce gage de confiance que nous accordons à la nouvelle dynamique engagée par l'État, je demande avec force et sans ambiguïté que les 550 millions d'euros qu'il a mobilisés soient intégralement affectés à la desserte FTTH des dernières zones d'initiative publique de notre territoire, qui sont les plus coûteuses à réaliser. Je parle bien de la « desserte », ce qui, techniquement et réglementairement, a tout son sens. Je soutiens également la volonté de l'État d'expérimenter un dispositif de financement des raccordements non standards au FTTH en zone publique : il est en effet incompréhensible pour certains de nos concitoyens

En tant que sénateur et président de l'Observatoire national de la présence postale, je me permets d'appeler votre attention sur la mission d'aménagement du territoire de La Poste, qui est bien souvent le dernier réseau présent dans les territoires. Le maillage d'au moins 17 000 points de contact, prévus par la loi et répartis sur tout le territoire, est garanti dans les zones urbaines et les zones rurales, dans les territoires périurbains, dans les zones de montagne et en outre-mer. mission impose à La Poste une norme d'accessibilité dont le respect est assuré, chaque année, par les commissions départementales de présence postale territoriale. C'est également dans le cadre de cette mission que La Poste peut adapter sa présence agences postales communales, relais commerçants, guichets France services, équipements numériques, accompagnements des fragilités sociales ont ainsi pu voir le jour. Ce n'est pas aux élus de terrain que j'apprendrai qu'à travers La Poste, c'est tout le dynamisme économique et social de la commune qui est en jeu.

Grâce au fonds postal national de péréquation territoriale qui finance la mission d'aménagement du territoire, les élus ont pu apporter des réponses concrètes. Autant d'actions nécessaires pour combattre la fracture numérique qui risquent de ne plus pouvoir être menées, si l'État ne respecte pas les engagements de financement

Le contrat encadrant la mission est signé par l'État, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité et La Poste. Les projets qui sont financés par le fonds postal de péréquation sont votés par les élus des commissions départementales de présence postale territoriale.

finances. Afin de financer le coût que représente sa mission d'intérêt général, La Poste bénéficie d'un allégement de fiscalité locale, dont le montant abonde le fonds postal de péréquation. Le taux des abattements appliqués aux bases de contribution économique territoriale et de taxe foncière est arrêté, chaque année, par décret, la CVAE représentant pas loin de 80 % de la base d'abattement alimentant le fonds.

Les commissions départementales de présence postale territoriale, composées d'élus locaux, n'auront plus de moyens à leur disposition et se verront privées de leur rôle. Elles deviendront des chambres d'enregistrement et de répartition de dépenses obligatoires.

cohérence, mes chers collègues ! En tant qu'élus, nous nous battons localement pour que La Poste reste dans nos quartiers et nos villages. Aujourd'hui, la question de sa présence et de son activité dans les territoires se pose à nous, en tant que législateurs, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. C'est pourquoi je vous invite à voter en faveur des amendements que j'ai déposés avec certains de nos collègues, afin de garantir le financement de la mission de service public d'aménagement du territoire de La Poste. Sous cette réserve, notre groupe votera les crédits de cette mission. La parole

C'est une garantie de qualité pour notre débat. Je vous répondrai en mettant en exergue trois objectifs fondamentaux de notre action. Le premier objectif de notre action, c'est de renforcer le soutien au commerce, à l'artisanat et aux territoires. La crise sanitaire est une épreuve pour nos commerçants, nos restaurateurs, nos artisans ou encore nos indépendants. Beaucoup d'efforts leur ont été demandés et nous en sommes pleinement conscients. Je veux d'abord les remercier de tous ces efforts consentis. Je comprends combien il est difficile de ne pas être autorisé à travailler tant qu'indépendant, on a engagé toutes ses économies, mis toute son énergie et fait des sacrifices immenses pour développer son activité. Face à ces difficultés, notre politique est très claire

Cette volonté de soutien aux commerces et de revitalisation de nos centres-villes se traduit également dans la mission « Économie » et les programmes déjà mis en place par le Gouvernement. Je pense, notamment, à la mise en oeuvre du programme « Action coeur de ville », qui comprend un axe dédié au développement économique pour soutenir le commerce de proximité et l'artisanat.

Le plan de relance prévoit par ailleurs 60 millions d'euros pour la création d'un fonds de déficit d'opérations d'aménagement commercial. Ainsi, et pour répondre aux questions soulevées par les rapporteurs spéciaux, nous mobilisons des moyens à la hauteur des enjeux. Le soutien à l'artisanat est également au coeur de nos préoccupations-

Nous inscrivons ainsi au projet de loi de finances pour 2021 la suppression sur trois ans de la majoration de la base taxable de 25 % pour les indépendants non adhérents d'un organisme de gestion. C'était une demande des professionnels, Le plan de soutien en faveur du commerce de proximité, de l'artisanat et des indépendants du 29 juin 2020, ainsi que le plan de relance amplifient cette stratégie. Enfin, l'État soutient l'économie des territoires. Il n'y a pas de désengagement en la matière, mais nous modifions la répartition des Nous avons mis en place un portage par les collectivités des aides aux entreprises, permettant de clarifier la répartition des rôles entre l'État et les régions en matière de développement économique. Cette évolution, en lien avec la loi du 7 août 2015 portant Concernant l'État, nous assumons avoir mis fin à certains dispositifs qui s'avéraient peu opérationnels pour privilégier des outils plus efficaces. Afin de rendre plus lisibles les crédits budgétaires et le pilotage du soutien aux entreprises, le programme 134 ne porte plus d'aides individuelles.

Le troisième objectif de notre action, c'est de poursuivre les réformes, car elles ont fait leurs preuves. Nos choix en matière de soutien à l'export et de diplomatie économique nous ont permis de devenir la première destination pour les investissements directs étrangers en Europe. Il faut continuer. Concernant l'export et l'attractivité, nous avons inscrit des moyens destinés au développement international des entreprises, dans le cadre de démarches pluriannuelles engagées par l'État avec Business France et Bpifrance Assurance Export. Nous n'avons d'ailleurs pas